après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

la France a besoin de ses armées. Elle a besoin d'une défense forte, solide, moderne. Elle en a besoin face à des menaces violentes, diffuses, mouvantes, face à des ennemis indéterminés. Les Français ont besoin de leurs armées. Elles sont la garantie de leur sécurité, de leur liberté. Elles sont la garantie de notre capacité à être entendus et écoutés. Le monde dans lequel la France évolue a été décrit avec précision et lucidité lors des travaux de la revue stratégique. Nous en avions débattu dans cet hémicycle, et nous en avions partagé le constat, comme les conséquences. Le constat est celui d'un monde plus violent, où le terrorisme continue de frapper, où les États reprennent la course aux armements. Un monde où les puissances s'affirment par tous moyens, où les dictateurs gazent leur propre peuple. Un monde instable, où les pratiques changent et les ennemis n'ont parfois ni motivation ni visage, mais continuent de frapper par des actions terroristes toujours plus barbares, y compris sur notre sol. Face à ce monde, nous l'avions dit clairement, la France doit agir. agir en donnant à ses armées tous les moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions. Elle doit agir pour répondre à toutes les menaces, être capable d'intervenir sur tous les terrains face à tous les ennemis. agir en disposant d'une ambition forte et d'un objectif clair : donner à nos armées des moyens à la hauteur et bâtir un modèle d'armée complet et équilibré. Nous le devons à nos armées. Nous le devons aux Français. Ce projet de loi de programmation militaire c'est une réponse une réponse à l'appel de nos armées. Une réponse à la demande des Français. Une réponse aux menaces qui pèsent sur notre pays. La loi de programmation militaire 2019-2025 est la première loi en expansion depuis la fin de la guerre froide. C'est le début d'une remontée en puissance historique. En effet, ce n'est pas un projet de loi de programmation militaire ordinaire dont nous débattons aujourd'hui : ce sont les fondations solides d'armées modernes, prêtes, prêtes, équipées. Il nous fallait investir massivement dans les armées. C'est ce que fait ce projet de loi. Le cap fixé par le Président de la République ne pouvait être plus clair : 2 % de la richesse nationale française sera consacré à la défense d'ici à 2025. Dès l'année 2017, j'ai obtenu le dégel de 1,9 milliard d'euros pour notre défense, permettant ainsi de respecter le budget 2017. extérieures, les OPEX, ont été couverts en interministériel par des ressources supplémentaires pour le budget de la défense. Pour cette année, la loi de finances initiale pour 2018 marque la première marche de la remontée en puissance de nos armées, avec une augmentation de 1,8 milliard d'euros de son budget. Concrètement, après des années de baisse continue, l'effort de défense, en pourcentage du PIB, a remonté cette année. Cette remontée en puissance se poursuit et s'accélère dans le présent projet de loi : 295 milliards d'euros seront ainsi consacrés à la défense sur la période de la programmation. Certains craignent que ces moyens n'arrivent trop tard. Or, rien que sur la période 2019-2023, ce sont 198 milliards d'euros qui seront investis pour notre défense, soit 23 % de plus que sur la période couverte par la précédente loi de programmation militaire.

C'est un projet de loi solide, un projet de loi budgétairement sincère. Bien sûr, j'entends les craintes. Je pense au surcoût des OPEX et des missions intérieures. Le Président de la République l'a dit et répété, la provision pour les OPEX et les missions intérieures, bien trop faible ces dernières années, a été augmentée à 650 millions d'euros en 2018, pour être portée à 1,1 milliard d'euros Parallèlement, ce texte inscrit noir sur blanc que les surcoûts éventuels seront financés en interministériel. Avec cette hausse de la provision, nous atténuons donc l'incertitude dans laquelle se trouvait le ministère concernant les ressources disponibles pour financer les opérations extérieures, qui,, faisait peser un risque sur les crédits d'équipement, trop souvent mis à contribution pour couvrir les OPEX. Cette décision rend nos budgets plus sincères, comme cela avait été demandé à de nombreuses reprises sur les travées de cette assemblée.

Je connais aussi les doutes de certains sur le financement du service national universel. Le Président de la République l'a affirmé plusieurs fois

et la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a choisi de renforcer ces dispositions. Toutes les garanties sont donc Je pense, enfin, à l'actualisation de 2021. Elle aussi est une garantie, et non un sujet d'inquiétude. Elle est la garantie de la bonne exécution de la loi de programmation militaire, Elle est le gage que nous emploierons les bons moyens pour atteindre l'objectif de 2 % du PIB en 2025. Déterminer dès aujourd'hui les crédits postérieurs à 2023, c'est risquer de nous tromper, c'est risquer de sous-estimer l'effort nécessaire. Nous le savons, l'enfer est pavé de bonnes intentions. À cet égard, il serait préjudiciable à nos armées que nous manquions l'objectif que nous nous étions fixé, faute d'avoir anticipé parfaitement l'évolution de notre PIB. Cette actualisation en 2021 est donc une bonne chose. J'en veux pour preuve l'actualisation de la LPM précédente, qui a permis, en 2015, de réajuster les ressources à un niveau plus conforme aux besoins.

Je veux le dire à tous : le rendez-vous de 2021 est une bonne chose, une garantie pour l'exécution de ce texte, une garantie pour les 2 %. 2 %. Je voulais vous dire que je comprends les craintes, mais aussi votre vigilance. Comment ne pas les comprendre après que tant de sacrifices ont été demandés à notre défense ? Je sais quel a été le rôle clé du Sénat, en soutien constant de nos armées quand les moyens n'étaient pas au rendez-vous. Depuis longtemps, et au cours de la dernière mandature en particulier, les sénateurs ont porté, en étroite collaboration avec Jean-Yves Le Drian, la défense d'un budget adéquat pour nos armées dans un contexte budgétaire particulièrement contraint. Ils ont contribué à préserver ce qui devait l'être, avec des ressources inférieures aux besoins, compte tenu du niveau très élevé d'engagement de nos armées. Cela a permis de répondre aux exigences de la défense nationale et aux besoins des femmes et des hommes qui servent pour notre pays. Je tenais à le souligner tout particulièrement. Ce combat, mesdames, messieurs les sénateurs, vous l'avez poursuivi depuis un an. Monsieur le président Cambon, vous avez su prendre la mesure de l'importance de ce texte pour notre défense comme pour nos militaires. Vous avez su le porter au-delà des débats politiciens, pour travailler dans le seul intérêt de notre défense et de nos armées. Avec vous, c'est toute une commission qui s'est emparée de cette loi de programmation militaire. Je tenais à rendre un hommage tout particulier au travail mené en commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, un travail qui a montré votre engagement pour notre défense, qui a montré une volonté, votre volonté d'enrichir ce texte pour le bien de nos armées. Je crois profondément au travail parlementaire et à la coconstruction législative. C'est pourquoi, dans le débat qui s'annonce, je serai particulièrement attentive aux changements réalisés lors de l'examen du texte en commission. Je ne vais pas égrener les thèmes il faut garder un peu de suspense pour la discussion des articles -, mais je peux d'ores et déjà vous dire que je soutiens une bonne partie des apports de la commission, sur le volet programmatique comme sur le volet normatif.

Ils permettront d'inverser résolument la courbe des recrutements et de nous préparer aux conflits du futur. Nous avons donc les moyens. La question qui se pose est celle de leur répartition. Ce projet de loi s'articule autour de quatre grands axes, dont chacun de réparer les carences du passé et de préparer l'avenir de nos armées. Le premier choix de cette loi de programmation militaire, c'est de se placer à hauteur d'homme. Les précédents textes ont toujours placé en leur coeur les gros équipements ; celui-ci tient d'abord compte de celles et ceux qui se battent pour nous. C'est un choix que j'assume, que je revendique et dont je suis fière. Depuis des années, les premières coupes budgétaires des gouvernements se faisaient au détriment des petits équipements. On enlevait donc à nos forces d'abord ce qui était le plus nécessaire à leur quotidien. Nous ne pouvions plus le tolérer. C'est pourquoi ce projet de loi prévoit la livraison de 55 000 gilets pare-balles dernier standard, dont 25 000 dès l'année prochaine.

Ce projet de loi de programmation militaire, ce sont aussi de nouveaux droits civiques. Il autorise en effet les militaires à siéger dans les conseils municipaux de certaines communes. C'est une mesure de justice. Il ne s'agit pas de faire de la politique, mais de laisser à des militaires les moyens d'un engagement local et de permettre à toutes les communes- surtout les plus petites -de bénéficier de tous les talents, de toutes les bonnes volontés. ce projet de loi amplifie les mesures prévues dans le plan Famille, dont la plupart des dispositions entreront en vigueur dès cette année. Très concrètement, cela signifie du wifi, des places en crèche, des logements supplémentaires et des affectations connues plus tôt Ce projet de loi donne de meilleures conditions de vie et d'exercice à nos militaires et à nos civils. Il maintient l'envie de s'engager et permet de continuer à vivre son engagement tout au long de sa vie. j'aimerais citer une mesure emblématique : ce texte permettra à tous les militaires, femmes et hommes, en congé pour convenance personnelle afin d'élever leur enfant,

le succès de nos opérations, ce texte prévoit un renouvellement majeur de nos capacités opérationnelles et une augmentation des cibles les plus stratégiques. Nous aurons sans doute l'occasion, au cours du débat, de revenir sur ces cibles et sur l'avancée des principaux programmes. Je ne vais donc pas me lancer dans un inventaire à la Prévert.

Certains de nos matériels sont usés, vieillissants, parfois même inadaptés. Leur renouvellement n'est donc pas une option, c'est un impératif absolu. Réparer et préparer : je l'ai déjà dit, c'est l'une des lignes fondatrices de ce texte. Contrairement aux précédentes lois de programmation militaire, ce projet ne procède à aucune annulation de programme ou renégociation massive de contrats, compte tenu des dernières exécutions qui ont été conformes aux ressources annoncées. Nous allons donc, pour les trois armées, réparer les déficits capacitaires, relancer les programmes et les accélérer. Pour l'armée de terre, nous allons accélérer le programme Scorpion. Par ailleurs, 50 % des nouveaux blindés médians auront été livrés d'ici à 2025. La marine bénéficiera de nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque, de nouvelles frégates, de patrouilleurs modernes en plus grand nombre.

Armée de terre, marine, armée de l'air : aucune impasse n'a été faite. Les trois armées voient leurs capacités renforcées, modernisées et accrues pour les plus stratégiques.

C'est le respect de l'engagement du Président de la République et c'est un choix que je revendique, car il n'est pas question de jouer aux dés avec le coeur de la souveraineté de notre nation ni de baisser la garde, alors que notre environnement stratégique se détériore un peu plus chaque jour. Le troisième fondement de cette loi de programmation militaire, c'est justement la garantie de l'autonomie stratégique de la France. C'est s'assurer que la voix de la France sera toujours entendue, écoutée, respectée. C'est s'assurer que nous serons capables de l'emporter, toujours, partout et tout le temps. Ce projet de loi de programmation militaire prend donc acte de la métamorphose des conflits actuels. Il nous faut anticiper mieux, prévoir, savoir. C'est pourquoi cette LPM accorde des moyens exceptionnels au renseignement, avec 1 500 nouveaux postes et 4,6 milliards d'euros d'investissements pour ses équipements. Ce projet de loi prend aussi le tournant et la mesure des enjeux de cyberdéfense, puisque nous investirons 1,6 milliard d'euros pour la lutte dans le cyberespace et que nous recruterons 1 000 cybercombattants supplémentaires d'ici à 2025. La France a la plus grande armée d'Europe. Avec ce texte, elle conforte sa place. Je dirais même plus : la France assume sa place. Elle en assume les forces, comme les responsabilités, au premier rang desquelles celle de fédérer, de faire le choix des projets ambitieux, des coopérations à grande échelle plutôt que des succès étriqués. Nous devrons nous tourner vers nos alliés, en particulier européens, et chercher des projets fédérateurs, stratégiques. Je pense à notre politique spatiale, à notre groupe aéronaval ou à la défense aérienne élargie. Nos voisins européens sont confrontés aux mêmes menaces, affrontent les mêmes dangers et partagent les mêmes constats

Nous la construirons autour d'opérations communes, autour de projets concrets. Il ne s'agit pas d'un pari sans fondement, d'une déclaration d'intention sans rien derrière : les lignes bougent. Je pense à l'initiative européenne d'intervention, je pense à la coopération structurée permanente. Je pense aussi à cet accord historique que j'ai signé, voilà quelques semaines, avec mon homologue allemande, pour le système de combat aérien futur. Nos deux États se sont mis d'accord pour travailler ensemble sur un projet structurant pour notre défense aérienne. C'est donc le début d'opportunités exceptionnelles pour l'Europe et pour notre industrie de défense. Enfin, Enfin, le dernier axe de cette LPM 2019-2025 que j'évoquerai est l'innovation. C'est une orientation à laquelle je tiens tout particulièrement et c'est, je crois, une nécessité pour conserver notre supériorité opérationnelle. On ne se prépare pas aux conflits du XXI siècle comme à une guerre de tranchées. S'accrocher coûte que coûte aux équipements ou aux doctrines actuels sans anticiper le futur, c'est comme se retrancher derrière la ligne Maginot. Aussi, avec cette loi de programmation militaire 2019-2025, les armées font pleinement leur entrée dans la modernité. Le numérique est présent partout. Nous devons donc l'intégrer dans toutes nos technologies et tous nos modes de combat. Nous devons nous emparer de la recherche, nous placer à sa pointe et créer des ponts entre l'économie civile et l'économie militaire. Ces enjeux sont déterminants pour nos armées. Ils le sont aussi pour notre économie, pour les 200 000 emplois de l'industrie de défense, pour les 4 000 PME de la base industrielle et technologique de défense. Ils le sont également pour les start-up, pour les inventions qui feront, demain, notre quotidien. La recherche militaire a déjà inventé internet, le pneu et le GPS, pourquoi s'arrêterait-elle maintenant ? Et pourquoi ces inventions seraient-elles l'apanage des Anglo-Saxons ? Ce texte nous donne les moyens de réussir. Nous augmenterons les moyens des études et de l'innovation en les portant de 730 millions d'euros par an à 1 milliard d'euros dès 2022. Nous créerons une agence de l'innovation de défense. Nous prendrons le tournant des défis de demain, en investissant, par exemple, 100 millions d'euros par an dans l'intelligence artificielle. Avec ce projet de loi, nous préparons aussi l'avenir en engageant les phases préparatoires des grands programmes d'armement qui structureront l'avenir de nos armées 1,8 milliard d'euros par an en moyenne seront ainsi consacrés à ces études qui nous permettront de concevoir le char de combat du futur, le système de combat aérien futur, dont je parlais à l'instant, ou le successeur du porte-avions. L'innovation, c'est un mode de pensée, un état d'esprit. Avec cette LPM nous pourrons agir comme nous le souhaitons, briser les carcans, troubler les conservatismes.

Ces réformes sont nécessaires et je prends devant vous l'engagement ferme de les mener jusqu'au bout et de surveiller leur exécution- comme celle de la loi de programmation militaire elle-même. Mesdames, messieurs les sénateurs, l'attente de nos armées est forte. Les espoirs des femmes et des hommes qui servent notre pays sont immenses. Ce texte donne des moyens exceptionnels à notre défense : il permet de renouveler les équipements ; il donne l'opportunité de mieux vivre l'engagement militaire ; il rend nos armées plus fortes, plus prêtes à affronter les défis et les conflits de demain. Ne nous trompons pas de débat : aujourd'hui, nous ne discutons pas de l'exécution de la programmation- nous nous aurons ce débat, année après année, lors de l'examen des projets de loi de finances et des projets de loi de règlement. nous discutons d'une programmation qui redonne à notre outil de défense les moyens dont il a besoin pour accomplir l'ensemble de ses missions. Il s'agit de l'avenir de nos armées, de nos militaires, de notre défense. Alors, donnons-nous toutes les chances et bâtissons, ensemble, une défense forte, moderne et audacieuse. La parole

il était temps de mettre fin à vingt ans d'éreintement de nos armées. Face à ces menaces, chacun doit faire son devoir. Nos soldats font le leur, de manière admirable, jour après jour, nuit après nuit. Et je souhaite que mes premiers mots soient pour eux et qu'ils entendent l'hommage de notre assemblée des communes de France, qu'ils protègent à travers l'opération Sentinelle, jusqu'aux dunes de sable où, chaque jour, ils subissent les assauts du terrorisme et mettent leur vie en danger.

Votre LPM est indiscutablement marquée par une remontée des crédits et des effectifs, et nous nous en réjouissons. Faire son devoir, pour le Sénat, c'est évidemment soutenir l'inflexion positive que porte le Gouvernement, mais en contrôlant l'exécution de ce texte et le respect des engagements lourds que vous entendez prendre devant la représentation nationale aujourd'hui. Permettez-moi de saluer le travail de la commission que j'ai l'honneur de présider et qui a systématiquement privilégié l'intérêt national aux dépens, parfois, des sensibilités de chacun- que ses membres en trouvent ici l'expression de ma profonde reconnaissance -, pour lui permettre de garder le rayonnement que mes augustes prédécesseurs ont su lui donner. Après la « revue stratégique » qui a identifié les menaces, c'était avec impatience que la commission attendait ce projet de loi de programmation militaire.

Ce projet de loi comporte à l'évidence de très nombreux aspects positifs. Enfin les moyens remontent ! Après des années d'attrition,

Madame la ministre, vos priorités sont les nôtres : à « hauteur d'homme », régénération de nos moyens, favoriser l'innovation, mettre en avant la coopération La commission de la défense partage vos ambitions : il faut préserver l'autonomie stratégique, garder un modèle complet d'armée qui maintient la capacité à entrer en premier sur le champ.

pour nos soldats, les avions ravitailleurs et de transport, les patrouilleurs, notamment en outre-mer et, bien sûr, la rénovation programmée des deux composantes de nos forces de dissuasion nucléaire. Mais les parlementaires

Madame la ministre, nous avons de sérieux doutes sur cette hausse brutale en fin de période. Les deux tiers des équipements seront mis en oeuvre dans le dernier tiers de la LPM.

pour la défense, à la suite d'une décision dont tout le monde se souvient, en juillet dernier. Il eût été préférable de ne pas rater la première marche de ce difficile escalier.

nous manquons de visibilité sur le rythme des livraisons d'équipements ou sur les infrastructures, puisque nous devons nous contenter d'objectifs assez lointains- 2025 et 2030 -, sans les points de passage annuels. Cette question est d'autant plus cruciale que la LPM ne couvre qu'une partie des besoins. Il manque 1,5 milliard d'euros de crédits d'infrastructures. En 2025, 60 % des installations de la défense, nos casernes notamment, seront « dégradées ». De même, les recrutements nous paraissent trop faibles et trop lents : 450 recrutements chaque année pour des besoins que nous estimons à 2 500 par an. On est encore loin du compte. Je veux marquer ici notre inquiétude pour les services de soutien, et particulièrement le service de santé des armées, le SSA. Ils sont éreintés. Je rappelle que les personnels projetés du service de santé des armées sont à 200 % de de leur contrat opérationnel. Il en va de même du commissariat aux armées, pourtant essentiel à la qualité de vie en régiment. Certaines lacunes capacitaires ne seront pas résorbées en fin de programmation. L'« accélération » annoncée ne peut être mesurée précisément d'ici à 2022. Elle sera donc assez modeste. En 2025,

Votre programmation repose sur un autre pari, celui des coopérations capacitaires européennes. Vous avez bien évidemment raison, même si nous avons, ici encore, quelques observations à formuler. Notre partenaire naturel, c'est le Royaume-Uni. Or il est affaibli à la fois par le manque de moyens et par le Brexit. Nous avons besoin de travailler avec nos amis anglais, mais les conditions sont encore assez difficiles. Le partenariat avec l'Allemagne repose pour l'instant sur des affirmations politiques, certes volontaristes, qui butent sur une réalité industrielle et opérationnelle quelque peu différente.

De façon plus générale, que seront les coopérations européennes sans une préférence européenne pour l'achat des équipements ? Souvenons-nous de ce qui s'est passé en Pologne et aux Pays-Bas et qui se répétera peut-être demain dans des pays plus proches ... Espérons que le bon sens l'emporte.

pour que ce service national universel ne soit financé ni en crédits ni en personnels par les ressources de la programmation militaire. Faute de quoi, la LPM disparaîtrait. Le Président de la République l'a promis

Sur les OPEX, la commission a inclus dans le calcul de leur coût l'usure accélérée du matériel en opération. Le ministère des armées ne paiera pas plus que sa part dans le budget général. De même, notre commission a enfin fixé le principe d'un retour intégral aux armées des produits de cessions immobilières, soit la coquette somme de 500 millions d'euros sur la programmation. Quand le ministère de la défense vend un immeuble, l'argent de cette vente doit lui revenir. Le principe est assez simple.

La commission a aussi souhaité mieux protéger les droits des pensionnés et des invalides de guerre en réintroduisant, au sein du contentieux administratif, les spécificités des formations de jugement actuelles. S'agissant de la possibilité pour les militaires de se faire élire dans les communes, sujet qui nous a mobilisés un certain temps et reviendra sûrement en discussion au cours de la soirée, la la commission a souhaité porter à 30 000 habitants le plafond au-dessus duquel les militaires en activité ne pourront pas être conseillers communautaires. En effet, le plafond de 15 000 habitants réduisait singulièrement la portée de ce texte. également supprimé l'interdiction pour les militaires élus dans les communes de moins de 9 000 habitants de participer à l'élection sénatoriale. Ne faisons pas des militaires des conseillers municipaux de seconde classe ! Ils doivent pouvoir exercer leur rôle comme un élu normal. Enfin - c'est un point très important -, la commission a voulu accroître les pouvoirs de contrôle du Parlement, dans le droit fil du souhait du Président de la République, qui nous avait réunis à Versailles pour nous demander d'approfondir les procédures de contrôle parlementaire.

que de décevoir. Ne vous affolez pas devant la volonté d'un contrôle parlementaire. Mon illustrissime prédécesseur Georges Clemenceau expliquait de cette tribune que le contrôle parlementaire est indispensable au succès de l'action militaire du gouvernement. Bravo ! Méditons tous ensemble cette phrase.

Avec ces capacités nouvelles, la France pourra, mieux encore, accomplir sa vocation, celle d'une grande puissance qui, bien armée, sera plus efficace encore au service de la paix. La parole

Ce terme de réparation n'est pas neutre : il exprime votre sentiment sur les moyens de nos armées et sur la situation dont vous avez hérité. Les causes sont bien connues des moyens encore revus à la baisse par rapport à la période 2009-2014 et une activité opérationnelle dont la durée et l'intensité ont été bien supérieures aux prévisions affichées. C'est ce qui nous avait conduits à qualifier à plusieurs reprises le budget des armées d'insincère. C'est à l'aune de ce critère de sincérité que la commission des finances a examiné le texte que vous nous soumettez.

évoquée ; la fin des recettes exceptionnelles improbables ; et une meilleure prise en compte du soutien à l'exportation. Sur le plan des dépenses, l'effort est également incontestable création de 6 000 postes, amélioration de la condition militaire, crédits d'équipement majorés permettant le renouvellement de la dissuasion nucléaire, renouvellement de certains matériels, efforts en faveur des infrastructures et meilleur entretien programmé des matériels. Pour autant, peut-on qualifier cette LPM de totalement sincère au sens budgétaire du terme ? Des points de fragilité, qui sont autant de points de vigilance, méritent d'être relevés. Le premier, chacun l'a bien à l'esprit, c'est que le gros de l'effort est reporté à la législature suivante et au prochain quinquennat : les crédits des armées augmenteront ainsi de 1,7 milliard d'euros par an jusqu'en 2022 et de 3 milliards d'euros par an à partir de 2023. À charge pour vos successeurs de trouver Par ailleurs, si les besoins sont bien programmés jusqu'en 2025, les annuités 2024 et 2025 ne sont pas couvertes de manière ferme. La même logique est appliquée en matière d'effectifs : sur les 6 000 créations de postes prévues, 4 500 sont renvoyées à après 2022. La question du porte-avions est tout juste effleurée, alors qu'une décision devra être prise avant le terme de cette LPM si nous voulons être prêts pour la date de 2038. Le deuxième point de vigilance, et non le moindre, c'est que les contrats opérationnels assignés à nos armées sont pratiquement inchangés par rapport à ceux qui étaient inscrits dans la précédente LPM. Or ces derniers ont été très largement dépassés et rien ne laisse penser que notre engagement puisse diminuer dans les prochaines années, bien au contraire ! Cela signifie, les mêmes causes ayant les mêmes effets, que l'effort engagé permettra sans doute de stopper la dégradation de nos capacités, mais leur régénération n'aura véritablement lieu qu'au cours du prochain quinquennat. Le troisième point de vigilance, c'est que, à la différence de la précédente loi de programmation, ce texte ne prévoit pas de clause de sauvegarde en matière d'évolution des prix des carburants opérationnels, renvoyant à l'actualisation de 2021.

en particulier du A400M et du NH90, qui sont loin d'être acquises. À ce titre, si l'on peut se réjouir d'une volonté de coopération avec nos partenaires, notamment l'Allemagne, les questions de propriétés industrielles et d'autorisation d'exporter, qui ne relèvent pas des mêmes procédures dans nos deux pays, sont loin d'être réglées. Notre industrie et notre souveraineté nationale ne peuvent en faire les frais. Ces points de vigilance ont fait l'objet d'un travail approfondi entre la commission des affaires étrangères et de la défense, saisie au fond, et notre commission des finances, saisie pour avis. Les amendements que nous avons déposés et adoptés en commission ne remettent pas en cause la trajectoire budgétaire proposée par le Gouvernement, ni les priorités que vous avez définies.

Aussi ne comprendrions-nous pas que le Gouvernement, au Sénat, ou selon une technique maintenant bien éprouvée avec l'Assemblée nationale, les rejette tous, pour revenir au texte initial. Vous êtes attachée à rétablir et conforter le lien État-Nation. En entendant le Parlement, vous y contribuerez. La fonction régalienne dont vous avez la charge appelle au consensus. Nous y prendrons notre part en votant votre texte, mais vous devez aussi donner des garanties au Parlement que cette loi de programmation sera bien exécutée. Tel est l'état d'esprit dans lequel nous abordons ce texte. La parole

pour reprendre l'expression de M. le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Deux titres extraits du rapport pour avis de la commission des lois résument notre analyse. premier : « Soutenir les besoins des armées tout en assurant la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ». Notre pays a besoin d'une « remontée en puissance

avec la question européenne des valeurs, la conditionnalité des aides européennes en fonction de ces mêmes valeurs, et la montée des nationalismes un peu partout autour de nous. C'est dire, mes chers collègues, qu'il doit y avoir en toute matière place à une régulation en fonction du droit. L'efficacité militaire n'est pas étrangère aux valeurs démocratiques. Plus ce modèle est mis en cause - reconnaissons-le - aux niveaux mondial

nous ne le rejetons pas en bloc, nous l'estimons néanmoins insuffisant. De surcroît, nous affirmons qu'il agit en trompe-l'oeil, laissant croire qu'une hausse des budgets effacerait le reste des manquements en matière de politique étrangère et militaire du Gouvernement. Ce que nous affirmons depuis longtemps déjà, c'est que la France doit conserver, ou plutôt retrouver, son indépendance, afin que notre pays puisse avoir sa voix propre dans le concert des nations. Or force est de le constater, malgré certaines avancées dans ce qui ne reste qu'une projection, la réalité demeure bien éloignée de cet objectif. Sur le plan financier, le flou, qui n'a rien d'artistique, entourant le financement du budget des OPEX, d'ailleurs largement sous-évalué, n'est plus acceptable. Qui des armées ou de l'interministériel en assumera la charge ? Mystère ... À ce jeu de « la roulette de Bercy », nos armées sont perdantes, car les arbitrages se font au détriment des programmes d'équipements. Or rogner sur ces derniers, c'est jouer avec la vie de nos soldats. Sur le plan stratégique, nous ne voulons pas d'un alignement aveugle sur les positions des États-Unis. L'OTAN exerce une tutelle trop forte sur la politique de défense française. De ce point de vue, notre réintégration fut une erreur, et elle le reste. Sur le plan militaire, nous sommes isolés au Mali et notre armée s'y use. Sur le dossier syrien, notre intérêt n'est pas d'affaiblir le régime d'Assad, que nous estimons être un rempart contre le terrorisme islamique, malgré vos affirmations, madame le ministre. Sur le plan industriel, ensuite, nous dénonçons la stratégie issue tout droit du « macronisme », que l'éphémère ministre de la défense Sylvie Goulard avait décrit en ces termes : « Si nous voulons faire l'Europe de la défense, il va il va y avoir des restructurations à opérer, à faire des choix, des choix de compatibilité et, à terme, [des choix] qui pourront passer dans un premier temps aboutissant à privilégier des consortiums dans lesquels les Français ne sont pas toujours leaders Vous avez bradé STX à Fincantieri pour moins de 80 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est Naval Group qui est menacé. Si nous n'avons rien, bien au contraire, contre des accords bilatéraux, ceux-ci doivent reposer sur des intérêts communs. Cela ne fonctionne pas avec nos partenaires allemands, qui, eux, agissent pour préserver leurs propres intérêts. Comment les en blâmer ? Nous dénonçons un changement amorcé depuis déjà plusieurs années, celui d'une dépendance mutuelle avec nos partenaires européens, qui se traduira à terme par l'abandon de notre système de défense nationale. Ce que vous qualifiez d'« efforts financiers » reste cruellement insuffisant. Les budgets annuels de votre LPM sont au-dessous des efforts financiers allemands et britanniques et ne tendront vers les 2 % du PIB qu'en 2025. Il ne peut exister de diplomatie indépendante sans une armée indépendante, sans une industrie nationale d'armement indépendante, sans un gouvernement indépendant. À la vue courtermiste d'un banquier d'affaires au regard figé sur sa comptabilité, nous préférons quant à nous la vision nationale et historique de souveraineté. C'est l'honneur et l'intérêt de la France de maintenir, comme elle l'a fait tout au long de son histoire, en tout cas jusqu'à un passé récent, une voix souveraine et non alignée. Nous avons les outils, nous avons l'intelligence, nous avons l'expérience, nous avons les soldats prêts au sacrifice de leur vie, pour que vive la France, et, pourtant, vous vous appliquez à les démanteler un à un. Au nom de la France, de son armée et de ses soldats, nous ne pouvons l'accepter.

Quand l'espoir naît d'un côté, il s'évanouit de l'autre. Quand la Corée du Nord semble faire un pas sur le dossier nucléaire, l'accord de Vienne avec l'Iran est fragilisé ! Quand Daech perd du terrain en Irak et en Syrie, l'organisation se dissémine et frappe ailleurs, en Afghanistan ou en Indonésie ! Le Yémen s'enfonce dans la crise et la bande de Gaza s'enflamme s'enflamme de nouveau. Aussi, dans ce contexte de menaces persistantes, notre pays doit non seulement maintenir, mais aussi renforcer son modèle d'armée. J'ajoute que, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, la France en a le devoir. Le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 affiche une ambition chiffrée, celle de porter l'effort de défense à 2 % du PIB d'ici à 2025. C'est un objectif qui est largement consensuel

est le bienvenu, car nous savons combien la programmation a été malmenée par le passé. Elle a souvent fait l'objet de quelques « ficelles », qui ont entamé la sincérité budgétaire de la mission « Défense Je pense à l'usage abusif de recettes exceptionnelles, à la pratique du « gel » budgétaire ou encore, s'agissant des équipements, au recours aux décalages calendaires ou à la réduction des cibles. S'agissant de l'avenir, une meilleure sécurisation des recettes opérée ici et là dans ce projet de loi permettra peut-être d'éviter certains écueils. En tout état de cause, les moyens augmenteront sur toute la durée de la programmation, même si l'on peut regretter que l'accélération se fasse seulement à partir de 2022, avec tous les aléas économiques ou politiques que l'on pourrait par avance imaginer. du RDSE approuve en tout cas l'objectif à terme, d'autant que nous savons qu'il garantira aussi notre crédibilité au sein de l'Union européenne. C'est un fait, la sortie du Royaume-Uni, grande puissance militaire, alourdira notre responsabilité au sein de la politique de sécurité et de défense commune. Vous l'avez dit, madame la ministre,

Lecointre. Il s'agit aussi de préparer l'armée aux défis futurs, qui sont nombreux, avec les nouveaux lieux de confrontations que sont l'espace exoatmosphérique ou le cyberespace. Je m'arrêterai un instant sur la cybersécurité. L'ANSSI a dressé pour 2017 un bilan vraiment alarmant : plus de 2 000 signalements d'événements de sécurité numérique ont été détectés, dont 20 incidents majeurs. Il semblerait en outre que la multiplication des épisodes s'accompagne d'outils de plus en plus sophistiqués et dévastateurs.

sur les 6 000 emplois nouveaux créés, d'en affecter 1 500 à la cyberdéfense. Par ailleurs, sur le plan normatif, la cyberdéfense est également visée au travers des mesures prévues au chapitre L'amélioration des capacités de détection des cyberattaques, avec l'intervention renforcée de l'ANSSI sous le contrôle de l'ARCEP, ou encore le bénéfice du régime d'« excuse pénale » des militaires pour les cybercombattants sont des mesures qui vont dans le bon sens. notre armée, vous l'avez dit, madame la ministre, la moderniser, innover, c'est aussi la doter rapidement des nouveaux équipements indispensables sur le terrain, en particulier en OPEX. Je pense tout particulièrement aux drones, qui sont aujourd'hui au centre de tous les dispositifs opérationnels. Nous savons que l'armée ne peut plus s'en passer et que l'ennemi, même non étatique, utilise depuis quelques années déjà cette technologie, certes à petite échelle. On l'a vu dans la bataille de Mossoul, Daech utilisait contre nos militaires des mini-drones piégés.

Tout doit être fait pour qu'ils exercent leur fonction dans les meilleures conditions, car ils honorent la France. Leur engagement est pour nous une forme d'orgueil.

mes chers collègues, ce projet de loi de programmation militaire constitue pour le Sénat un rendez-vous majeur, puisqu'il s'agit de débattre et de voter l'orientation générale de notre défense et l'effort financier qui doit la soutenir, au cours de la période 2019-2025. Vous l'avez dit, madame la ministre, ce projet de loi donne à l'armée les moyens de son ambition. Notre budget de la défense est passé de 6,2 % de 6,2 % du PIB en 1962 à 1,54 % du PIB en 2014. Au lendemain du choc du 13 novembre 2015, de l'intervention Chammal dans l'espace assyrien dans l'espace assyrien et à l'heure du renforcement de notre présence au Sahel, l'érosion constante de nos crédits n'est plus acceptable. Je voudrais donc saluer votre détermination à tout mettre en oeuvre pour redonner à notre défense les moyens d'affronter les menaces auxquelles nous devons faire face et pour préparer nos armées aux défis de demain, en portant l'engagement du Président de la République d'atteindre progressivement un effort de défense représentant 2 % du PIB en 2025. Pour y parvenir, ce projet de loi de programmation militaire prévoit une hausse annuelle de 1,7 milliard d'euros par an jusqu'en 2022, soit de 5 % par an,

Il prend enfin en compte nos besoins et les besoins de nos soldats. Pour ce faire, il rompt avec la tendance de ces dernières années de réduction des effectifs. Après les 60 000 suppressions de postes dans les armées françaises entre 2005 et 2015, il est plus que louable que cette programmation vienne apporter un peu d'oxygène à nos armées, en prévoyant 6 000 postes supplémentaires d'ici à 2025, pour porter à cet horizon les effectifs à 275 000 personnes. Entre 2019 et 2023, il est ainsi prévu d'augmenter de 14 % les dépenses liées aux conditions de travail et de vie du militaire. Je me félicite, la ministre, de ce choix de conférer une place prioritaire à l'amélioration de la vie professionnelle et personnelle de nos soldats, alors même que 400 millions d'euros avaient déjà été consacrés au bien-être des familles

ambitions consiste à adapter notre outil de défense aux évolutions rapides du contexte géopolitique. À cet égard, il est important de tenir compte de l'ouverture de nouvelles perspectives en matière de coopération européenne de développement des armes et des technologies de défense conjointe. Comme l'a rappelé le Président de la République lors de ses voeux aux armées, « il ne s'agit pas de dupliquer ou de concurrencer l'OTAN, mais de réunir les conditions de l'autonomie stratégique de l'Europe ». C'est en ce sens que la décision de 25 pays de l'Union européenne de lancer une coopération militaire inédite, afin de développer en commun des équipements et des armements, mais aussi de faciliter les opérations extérieures menées, est une décision historique. De ce point de vue, je me félicite des avancées actées à la fin du mois d'avril à Berlin s'agissant de la coopération franco-allemande dans l'aéronautique, sur le système de combat aérien futur. La deuxième ambition véhiculée par ce projet de loi est de permettre à la France de continuer à assumer les responsabilités particulières qui sont les siennes en matière de sécurité internationale. Ces obligations entraînent des exigences lourdes : intervenir, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et membre de l'OTAN, dans le règlement de crises hors d'Europe, notamment en Afrique et au Proche-Orient. Les armées françaises seront capables de s'engager dans la durée et simultanément sur trois théâtres d'opérations ; de ce fait, la provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures, qui était jusqu'à présent toujours sous-estimée, est rehaussée. C'est là un choix cohérent et bienvenu. En outre, troisième ambition, ce projet de loi vise à poursuivre la modernisation de notre outil de défense dans un cadre financièrement crédible. crédible. Une enveloppe totale de près de 173 milliards d'euros est consacrée aux équipements et à leur entretien. Le texte accélère leur modernisation, tout en augmentant le nombre de certains équipements prioritaires. Par ailleurs, face à la course internationale au réarmement atomique, des travaux de renouvellement des deux composantes, navale et aérienne, de la dissuasion nucléaire seront engagés au cours de ce quinquennat, pour un budget de 37 milliards d'euros entre 2019 et 2025.

Plusieurs modifications et enrichissements ont été apportés lors de l'examen de ce texte en commission, parmi lesquels un point en particulier nous alerte, à savoir celui qui concerne la délégation parlementaire au renseignement. Mais nous aurons l'occasion, au cours de la discussion de ce texte, d'en débattre plus avant- je n'en doute pas.

programmation militaire dans un contexte géopolitique mondial où les conflits n'ont jamais été aussi nombreux. Nous faisons face à des guerres par procuration, des résolutions de l'ONU bafouées, des ingérences militaires multiples, des milliers de morts. Nos forces armées n'ont jamais été aussi mobilisées que ces dernières années. Toutes les opérations menées ont certes montré la puissance militaire de la France, mais aussi ses limites et ses insuffisances. Répondre aux difficultés du maintien en condition

Le texte prévoit une augmentation du budget à hauteur de 2 % du PIB. Cet objectif, décidé lors du sommet de l'OTAN de 2014, m'interroge. Sera-t-il suffisant ou insuffisant, alors même que le Gouvernement entend rogner partout ailleurs le budget de l'État ? Cela nous interpelle d'autant plus qu'une part non négligeable de ces moyens est mise en oeuvre dans le cadre du plan de modernisation nucléaire : 25 milliards d'euros jusqu'en 2023

Mes chers collègues, c'est démesuré ! Nous sommes loin de la lutte contre la prolifération et pour la diminution des armes nucléaires, ambition pourtant inscrite dans le traité de non-prolifération.

Madame la ministre, je connais et j'apprécie votre préoccupation concernant la sécurité de nos militaires- vous l'avez de

des troupes françaises à entrer les premières sur un terrain d'opérations extérieures et la sécurité des soldats reposent sur le service de santé des armées,

permettront de les augmenter, comme vous l'avez souhaité, afin de tenir compte de l'usure qu'a subie ce service ces dernières années.

d'un côté, un premier groupe d'États souhaite agir dans le cadre de l'ONU ; de l'autre côté, un second groupe d'États, actant des blocages réels des Nations unies, préférera s'affranchir de l'Organisation plutôt que de mener la réforme Certes, le droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité contraint trop souvent de nombreux pays à outrepasser les décisions de l'ONU- nous l'avons Mais l'alignement de plus en plus fort de la France sur les États-Unis par le biais de l'OTAN pousse notre pays dans le second groupe d'États, ce que nous condamnons vivement. Face à l'OTAN, nous est proposée dans cette LPM la réalisation d'une défense au niveau européen. Mais cette Europe de la défense se construira-t-elle en parallèle de l'OTAN ou en remplacement de celle-ci ? Cette question nous semble très importante. ailleurs, la question du développement toujours plus grand du commerce des armes, qui représente déjà 30 % de la production. Malheureusement, cette LPM s'inscrit dans la continuité d'une politique visant à rechercher l'équilibre de la balance commerciale par l'exportation d'armes. Permettez-moi de citer quelqu'un que vous admirez tous, ici, à savoir Ban Ki-moon, qui alertait sur la nécessité que « les États parties prenantes du traité sur le commerce des armes montrent l'exemple en contrôlant l'approvisionnement en armes d'acteurs qui pourraient les utiliser en infraction au droit international humanitaire. » Madame la ministre, je vous invite à suivre, avec autant de célérité que sur d'autres sujets, la position du Parlement européen, qui consiste à refuser l'exportation s'il existe un risque manifeste que la vente d'armes serve à commettre des violations graves du droit humain. : celui du Yémen, où des armes françaises ont été utilisées, et sont peut-être toujours utilisées, contre la population civile depuis des années. N'oublions jamais que les armes causent des souffrances immenses et multiplient les risques d'un embrasement général. Mes chers collègues, le tableau n'est toutefois pas totalement sombre. Ainsi, je me félicite des efforts faits en matière de recrutements sous statut. La prise en charge des réservistes reste perfectible, mais va dans le bon sens, tout comme le renforcement du maintien en condition opérationnelle et des garanties en termes de matériels individuels et de zones d'entraînement. Malgré ces améliorations, que nous avions souhaitées et qui étaient attendues par nos forces armées, nous déplorons le renforcement de l'arme nucléaire, qui va bien au-delà, selon nous, de la simple dissuasion, ainsi que les nouveaux accords avec l'OTAN.

madame la ministre, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord avoir une pensée pour les femmes et les hommes engagés dans les missions qui leur sont confiées en France et dans le monde pour assurer notre sécurité, saluer l'ensemble de nos forces armées, rendre hommage aux blessés et à ceux qui ont perdu la vie au service de notre pays. J'ai une pensée particulière pour toutes les femmes qui font de notre armée la plus féminisée d'Europe après l'armée Cette LPM s'inscrit malheureusement dans un contexte sécuritaire sous tensions : tensions internes, puisque la France reste sous une menace terroriste constante- les événements du 12 mai dernier dans le quartier de l'Opéra, à Paris, l'ont une nouvelle fois tensions externes liées à cette menace terroriste, mais également à beaucoup d'autres : la piraterie, le retour des États-puissances, l'effondrement de certains États, les conséquences du réchauffement climatique. Devant ces menaces, les moyens des forces armées doivent non seulement être consolidés, mais également relevés. Les différentes opérations militaires en cours appellent une progression du budget, afin de permettre à nos soldats de réaliser leurs missions dans les meilleures conditions de sécurité possible. Ainsi, il faut renforcer et moderniser les équipements et les installations de nos armées. Cela sera réalisable grâce à la présence sur nos territoires d'un tissu de dix grands groupes industriels et de près de 4 000 PME. Cette industrie de défense est un fleuron national qui tire l'ensemble de notre économie vers le haut, notamment par les emplois créés qui ne sont pas délocalisables. Maintenir notre puissance et nos capacités d'action, c'est aussi garantir que notre industrie de défense continue d'être un secteur clé de notre économie. Le volontarisme affiché par le Gouvernement devrait permettre aux industriels de la défense de produire davantage. Mais il ne faudrait pas que la planification 2019-2025, dont la part la plus importante des dépenses interviendra après 2022, reste modeste en début de programmation et nous mette en position d'infériorité dans le paysage de la Base industrielle et technologique de défense en cours de composition. La Direction générale de l'armement pourrait être tentée d'être précautionneuse lors de la phase transitoire de relèvement du niveau des autorisations d'engagement, grippant ainsi le système, et notamment les carnets de commandes des industriels. Cette LPM présente des perspectives positives pour les forces armées, avec la confirmation d'une hausse des crédits et la volonté d'accélérer certains programmes pour chacune des trois armées

réside aussi dans la confirmation de l'intention politique de consolider notre autonomie stratégique tout en renforçant nos partenariats au sein du continent européen. C'est un des fils rouges du rapport annexé. Si l'intention est louable, il nous faudra demeurer prudents et réalistes sur la capacité collective des Européens à cheminer ensemble. Nos cultures militaires sont différentes et les analyses stratégiques, souvent divergentes, ce qui n'exclut évidemment pas des convergences. La prise de conscience est là - la coopération structurée permanente et la mise en place du Fonds européen en témoignent -, mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres, en matière de réalisations. Passé les annonces et l'excellente communication qui les entoure, je souhaite revenir sur un certain nombre de points qui sont, à ce stade, autant d'interrogations. Le premier est un constat cette loi de programmation militaire est la treizième, et ses orientations s'inscrivent dans une forme de continuité avec ce qui a été décidé par le président Hollande en 2015, quand avait été annoncée une remontée en puissance de notre défense par le gel de la baisse des effectifs et par la stabilisation des crédits. point concerne la trajectoire financière. Lors des nombreuses auditions menées au sein de notre commission, les militaires et les industriels ont unanimement salué l'augmentation des budgets et des effectifs inscrite dans la LPM 2019-2025. Cependant, derrière cette augmentation, les premiers doutes se font jour. Comme pour les ressources financières- cela a été dit avant moi -, sur les 6 000 emplois promis, trois sur quatre sont envisagés pour le prochain quinquennat. Et si leur fléchage vers les secteurs du renseignement et de la cyberdéfense ou vers la protection des points sensibles nous semble pertinent, ceux qui sont dédiés aux exportations nous interpellent. nous nous interrogeons sur les 400 postes fléchés prioritairement sur les exportations, alors que les moyens consacrés au recrutement, à la formation, à la santé, ne sont pas suffisants et mériteraient d'être

Troisième point d'inquiétude : cette LPM abrite en son sein de réelles fragilités, liées à une trajectoire budgétaire surprenante. Pour répondre aux ambitions affichées par le Gouvernement, l'effort reposera sur une trajectoire budgétaire dont la moitié sera réalisée après les élections de 2022. Or le budget alloué dépendra de la croissance future et de la situation des finances publiques. Néanmoins, les investissements militaires ne peuvent se faire au détriment d'autres domaines régaliens. Autre lacune : les infrastructures sont fragilisées par une répartition des crédits peu opportune. Il aurait fallu, là aussi, un effort plus régulier ; en l'état, comme l'a rappelé le président Cambon, à l'horizon 2025, 60 % des infrastructures de la défense seront dégradées, voire inutilisables. Concernant les équipements, les lacunes capacitaires ne seront pas résorbées d'ici à la fin de la programmation, et nombre d'entre eux n'auront pas pu être rénovés. Cette loi de programmation militaire, au budget important, contient donc plusieurs faiblesses que nous ne pouvons occulter et auxquelles nous serons attentifs chaque année lors du vote du budget. La commission a adopté la LPM en raison de la remontée en puissance des moyens annoncés pour sécuriser les ressources de nos armées. L'enjeu, pour nous, parlementaires, sera de nous assurer de la réalité de ces moyens et de contrôler la bonne application Grâce aux nombreux amendements portés notamment par les commissaires de la commission des affaires étrangères et par mes collègues du groupe socialiste et républicain, nous avons sanctuarisé les crédits de la LPM, affirmé le rôle du Parlement, renforcé le volet immobilier, simplifié les processus d'acquisition, préservé les droits des pensionnés et invalides de guerre, précisé les dispositions relatives aux incompatibilités liées à l'éligibilité des militaires en activité. La triste réalité est qu'aujourd'hui seule la moitié du matériel militaire est utilisable. De nombreux parcs d'équipements souffrent d'une faible disponibilité- je pense aux hélicoptères de type Gazelle ou aux véhicules terrestres de type VAB -en raison d'une maintenance déficiente, d'une usure accélérée engendrée par la multiplicité des engagements, ou, simplement, parce qu'ils sont trop vieux. nous avons adopté en commission des amendements visant à la modernisation des équipements de nos forces. Concernant l'innovation, la commission a permis un assouplissement du cadre juridique des achats d'équipements, pour permettre une diffusion plus rapide et moins coûteuse de l'innovation. Dans le domaine du renseignement, le texte issu de la commission nous semble garantir une meilleure association du Parlement dans son rôle de contrôle, pour un partage efficace des informations.

Nous avons aussi obtenu que soit garantie la constitutionnalité des mesures de la LPM en matière de cyberdéfense. Autre sujet d'importance la question de l'immobilier. Les commissaires socialistes ont fait adopter un amendement tendant à garantir un effort financier important en faveur de la politique immobilière jusqu'en 2023. Cela permettra l'amélioration des conditions d'exercice du métier, celle du logement des militaires et de leurs familles.

Enfin, je défendrai à titre personnel, avec certaines et certains de mes collègues, des amendements en faveur de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans nos armées. des amendements visant à consolider le service militaire volontaire et son ouverture à l'ensemble des jeunes Français, y compris ceux qui résident à l'étranger, ainsi que des amendements visant à accompagner nos PME. Nous avons abordé la LPM non pas comme un exercice purement comptable, mais comme un texte ayant vocation à protéger les Françaises et les Français. Embrassant les défis stratégiques et technologiques qui s'imposent à nous, les effets induits par les progrès technologiques qui y sont qui y sont dessinés pourront se traduire par des applications civiles- il est ici important de le rappeler, dans la mesure où l'effort financier de cette programmation militaire repose sur les contribuables. Contrairement à ce qui s'était passé pour la revue stratégique, nous sommes associés à l'élaboration de ce texte, ce qui nous permettra de jouer notre rôle de parlementaires. Nous soutenons l'augmentation des crédits et des effectifs contenue dans cette LPM. Nous saluons également l'ambition européenne de ce texte. Nous restons favorables à une réelle coopération militaire européenne jetant les bases d'une véritable autonomie stratégique. Nous serons donc à vos côtés, madame la ministre, pour faire en sorte que cette trajectoire budgétaire soit respectée et que les avancées européennes se concrétisent. La parole

Cet engagement est ambitieux- cela a été rappelé -, mais il est également nécessaire. Il est nécessaire pour faire face au spectre des menaces identifiées par la revue stratégique de 2017 la lutte contre le terrorisme, bien sûr, mais aussi le retour de la compétition stratégique, la complexité croissante des armements et l'émergence de nouveaux espaces de conflictualité, comme le cyberespace et l'espace exoatmosphérique. Il est nécessaire pour réparer les dégâts d'une décennie de déflation, qui a mis en péril notre modèle d'armée. Il est nécessaire pour que notre responsabilité de modernisation de la dissuasion nucléaire et de défense de nos intérêts nationaux en tous lieux. Cette loi de programmation militaire doit faire converger enfin l'ambition et les moyens destinés à nos armées. Mais la question de sa soutenabilité se pose inévitablement : il faudra de la vigilance et de la ténacité politique pour la faire appliquer. L'exécution des précédentes lois de programmation militaire a montré que de bonnes intentions peinent parfois à se traduire dans les faits. Pour vous aider à réussir une telle traduction, madame la ministre, sous l'impulsion du président Christian Cambon,

évoquer maintenant la partie normative de la loi sous le prisme du programme 212, composante essentielle de cette loi de programmation militaire. En matière de politique immobilière, d'abord, vous avez fait un pas vers davantage de sincérité. Mais nous devons aller plus loin : il faut sécuriser le retour au ministère des armées de l'intégralité de ses produits immobiliers et aménager enfin la décote « Duflot », qui est une catastrophe financière pour ledit ministère, dont le le patrimoine est un véritable atout pour notre effort de défense. C'est une ressource essentielle. Il est temps de cesser de la brader. J'en viens aux ressources humaines. Le projet de loi prévoit une augmentation nette de 6 000 équivalents temps plein sur la durée de la programmation. C'est très en deçà des 50 000 emplois supprimés depuis 2008, mais les priorités des affectations, la cyberdéfense et le renseignement notamment, sont cohérentes. Le lancement d'un plan Famille a également été une heureuse décision. Nos soldats et leurs familles méritent alors que depuis dix ans ils subissent la dégradation de leurs conditions de vie, de travail et de sécurité, couplée à un engagement opérationnel toujours croissant. voulu, madame la ministre, mettre cette loi de programmation militaire « à hauteur d'homme ». L'accent a été mis sur les petits équipements, les infrastructures et le maintien en condition opérationnelle. La reconversion des militaires dans la fonction publique est facilitée ; les contraintes pesant sur l'éligibilité des militaires sont allégées. Je souhaite par ailleurs évoquer la reconnaissance due à nos vétérans et aux soldats morts en opération. des premiers, la réforme du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est une nécessité désormais reconnue, qui doit préserver la singularité du droit à réparation prévue par le code actuel. les seconds, nous souhaitons que le Gouvernement se penche enfin sérieusement sur la possibilité d'attribuer la mention « Mort pour la France » aux militaires déployés dans le cadre des opérations intérieures comme l'opération Sentinelle. Mon groupe déposera une proposition de loi en ce sens. Mes chers collègues, cette loi de programmation militaire était celle de la dernière chance pour un modèle d'armée au bord de la rupture. Plus encore, cette loi de programmation militaire est une composante du redressement national, tant il existe un pacte séculaire entre la grandeur de la France et la grandeur Sans méconnaître le chemin qu'il reste à parcourir, le groupe Les Indépendants votera en faveur de cette cinquième loi de programmation militaire, probablement la meilleure dont nous ayons eu à connaître depuis au moins vingt ans. Pour conclure, je souhaite féliciter et remercier chaleureusement l'équipe des collaborateurs de la commission des affaires étrangères, pour l'excellence de son travail de préparation de nos débats. Sa compétence est essentielle ... Très bien ! ... dans un moment où nous avons tous collectivement le privilège et la responsabilité de préparer notre pays à relever les défis de l'avenir et à affronter les tumultes du monde. La parole

madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, la loi de programmation militaire 2019-2025 intervient dans un contexte international tendu, tant aux pourtours de l'Union européenne qu'au Moyen-Orient ou en Asie. Nous sommes loin de la « fin de l'Histoire » annoncée par certains analystes il y a trente ans. Ces crises mal anticipées ont amené les armées à être engagées très au-delà de leurs contrats opérationnels, accélérant l'usure des matériels et des hommes, obérant les temps de repos ou de formation des personnels. Il apparaît peu probable qu'il en soit autrement demain, tant les foyers ardents de crise sont nombreux, les acteurs divers et imprévisibles. Se maintenir à ce niveau d'engagement me semble difficile ; aller au-delà serait hasardeux, voire dangereux. Personne ne peut dire de quoi demain sera fait ; c'est bien là la difficulté posée par cette LPM, qui renvoie l'essentiel de l'effort à des échéances plus lointaines. J'aborderai d'abord le programme 144, à propos duquel je m'attacherai au point, essentiel, des études amont. Mon appréciation, en la matière, est nuancée : le projet de loi- il faut le souligner -comporte un élément positif, à savoir l'augmentation des crédits d'études amont, mais celle-ci s'inscrit dans un contexte très flou. très flou. Cette hausse prévue de 37 % est bel et bien significative et correspond aux attentes de notre commission, exprimées l'année dernière, bien qu'on puisse toujours se demander si l'accélération des efforts de recherche des autres pays n'est pas plus forte et technologique de défense repose de façon importante sur ces crédits d'études amont. Ainsi, dans le cas de grands acteurs industriels présents dans le monde entier, ces crédits contribuent de façon importante à l'attractivité de notre pays

tenu, d'une part, du rôle qu'elles jouent dans l'innovation et, d'autre part, des difficultés d'accès aux financements bancaires, notamment liées aux règles de « compliance Madame la ministre, les banques préfèrent financer des applications pour mobiles que les PME de la défense ; c'est un problème sur lequel nous devrons nous pencher.

le déploiement du groupe aéronaval au Levant en a démontré toute la plus-value opérationnelle. Cela étant, compte tenu des délais, les études doivent être lancées au plus vite pour permettre au Président de la République de trancher à l'horizon 2020-2021.

Par ailleurs, dans un monde où la prolifération progresse de manière inquiétante, notre dissuasion, dans ses deux composantes, doit rester la garantie ultime de notre sécurité. Tout ajustement budgétaire inconsidéré entraînerait une perte de nos capacités opérationnelles, sur laquelle il serait quasi impossible de revenir ultérieurement. Sur les grands équipements, cette LPM prévoit des commandes permettant un renouvellement des moyens et un rattrapage, parfois lent, de certaines des lacunes capacitaires, comme pour les avions ravitailleurs, mais ne laisse guère de marge et renvoie à des échéances éloignées. Encore faut-il aussi espérer qu'il n'y ait pas de difficultés après l'entrée en service des équipements, comme ce fut le cas pour l'A400M ou certains véhicules des forces spéciales. Par ailleurs, je ne voudrais pas que, à trop vouloir montrer le principal, on en oublie l'accessoire, tout aussi indispensable. Ce renouvellement ne doit pas occulter la problématique des munitions, en particulier des munitions « complexes », pour lesquelles les dotations devront être suffisantes pour couvrir les opérations et l'entraînement. De même, si la LPM prévoit bien la modernisation des avions de patrouille maritime, il conviendra d'éviter les tensions sur les bouées acoustiques, essentielles dans la lutte anti-sous-marine, notamment pour la surveillance de nos approches. Depuis plusieurs années, assurer pleinement notre souveraineté sur notre zone économique exclusive, ou ZEE, est devenu un défi. Les évolutions du parc de patrouilleurs étaient plus que nécessaires. Au regard des espaces considérables de ZEE à surveiller, les mailles du filet resteront larges. Imagine-t-on un seul camion de pompiers pour couvrir la superficie d'une région comme la Bretagne ou ma Normandie ? Madame la ministre, nous devons préserver nos intérêts économiques, lutter contre les prédations sur la ressource halieutique, le sable et les autres richesses du sous-sol, et peut-être également demain défendre de vive force nos territoires lointains. Les ressources humaines constituent un autre point favorable abordé par la loi de programmation. Beaucoup a été demandé aux personnels de la défense, dans un contexte de déflations massives et de recrudescence des engagements. Nous saluons tous ici leur dévouement. Ne plus avoir à acheter eux-mêmes certains de leurs effets, pouvoir prendre leurs congés ou réussir leur reconversion, ce sont autant d'attentes légitimes des militaires. En outre, ces derniers ne sont pas des citoyens de seconde zone. Par conséquent, il me semble nécessaire de ne pas poser d'incompatibilités trop restrictives entre leurs fonctions et certains mandats locaux. Dans cet avenir incertain, beaucoup d'espoirs sont placés dans la coopération européenne, qui permet mutualisation et économies, au moment où la sophistication des équipements tire les coûts vers le haut. Gardons-nous toutefois de tomber dans l'excès de confiance. Il faudra plus que des déclarations d'intention et des moyens comptés pour contrer les mastodontes de la défense que sont les entreprises américaines et la montée en puissance des pays émergents. Ce nouveau « paradigme » ne doit dissimuler ni les écueils ni les résultats parfois mitigés en matière de coopération européenne. La convergence des doctrines, l'harmonisation des expressions de besoins et l'alignement des calendriers opérationnels sont des conditions du succès des coopérations, mais se révèlent difficiles à obtenir. Il faudra aussi s'entendre jusque sur les mots, car, en matière d'industrie de défense, la France pense « défense », alors que l'Allemagne pense « industrie Dans un partenariat industriel, ces divergences d'appréciation peuvent conduire à de graves désillusions. Pour simplifier, l'Allemagne produit et vend, tandis que la France tire et paye ! Cette asymétrie n'est pas viable durablement. Au final, si les coopérations sont mal conduites, elles aboutissent à des retards et des surcoûts. Au-delà des rapprochements, de la coopération, c'est aussi vers davantage de solidarité entre Européens qu'il faudra tendre. Pour conclure, dans une époque marquée par une multiplication des tensions et du terrorisme, alors que les vastes espaces de plus en plus contestés sont à surveiller, nous avons besoin d'un outil militaire moderne et dimensionné pour assurer notre sécurité. Cette loi de programmation est une étape, certes, positive, mais de nombreuses incertitudes persistent. Il en faudra sans doute davantage pour aborder l'avenir plus sereinement. Au final, madame la ministre, j'espère que vous saurez entendre les observations du Sénat retenir ses propositions, dans l'intérêt même du monde combattant. La parole Madame la présidente, madame la ministre, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi de programmation militaire dont nous commençons l'examen ce jour marque la fin d'une décennie d'érosion qui a abouti à des pertes d'effectifs importantes. texte conjugue avec le nécessaire renouvellement des équipements des armées la volonté de maintenir notre pays comme l'un des acteurs majeurs en matière de défense, en prévoyant de doter nos armées de matériels au meilleur niveau technologique et en nombre suffisant. C'est donc une LPM de remontée en puissance, mais également de défis. En effet, elle doit, en alliant budget et stratégie, instituer, d'une part, la dissuasion en enjeu majeur et, d'autre part, assurer la protection de notre territoire national, dans un contexte de menace terroriste permanente et de retour d'une rhétorique de puissance à l'échelon international. Cette loi de programmation militaire couvre la période 2019-2025, avec deux séquences : une première, de 2019 à 2022, avec un budget en hausse annuelle de 1,7 milliard puis, une seconde, de 2023 à 2025, avec une augmentation du budget des armées qui atteindra 3 milliards d'euros par an. La trajectoire est ambitieuse, mais elle peut apparaître douteuse après 2022, pour des raisons politiques, mais également par l'absence de trajectoire financière pour les infrastructures et par le manque de visibilité concernant les échéances de livraison de matériel. En ce sens, notre groupe Union Centriste a souhaité déposer un amendement ayant pour objet d'inviter le Gouvernement à réaliser avant le 1 janvier 2021 une actualisation de la revue stratégique de défense et de sécurité nationale, afin d'évaluer les mutations stratégiques à la date de cette actualisation. Notre travail en commission nous a d'ores et déjà permis de revenir sur de nombreux sujets. Je pense notamment à la question de la durée d'autorisation d'absence octroyée aux salariés des entreprises de plus de 200 salariés au titre de leurs activités de réserve. À la quasi-unanimité, nous avons ramené ce congé à huit jours, contre les cinq qui sont actuellement en vigueur, et au lieu des dix jours souhaités par nos collègues députés. En effet, ce passage à dix jours n'a jamais été sollicité, ni par les réservistes eux-mêmes, ni par les associations qui les fédèrent, ni par le ministère des armées, ni par le secrétaire général de la Garde nationale. Notre commission a également réintroduit à l'article 32, au sein du contentieux administratif, les spécificités des formations de jugement actuelles, et a précisé à l'article 36 les conditions de détermination des pensions militaires d'invalidité. Notre groupe veillera pendant les débats à ce que les droits des blessés et pensionnés soient préservés.

Madame la ministre, j'insiste sur ce point : l'extension du SMV ou la naissance du SNU ne doivent en aucun cas se faire au détriment des moyens dévolus à la défense proprement dite et aux objectifs initiaux. Un certain nombre de rapports ont d'ailleurs été réalisés sur le sujet. Je souhaite enfin évoquer le pari des coopérations capacitaires européennes. Le rapport de la Cour des comptes sur la coopération européenne en matière d'armement publié en avril 2018 présente un bilan peu encourageant et souligne que « la plupart des grands programmes en cours ont rencontré des succès technologiques parfois remarquables, mais aucun n'a atteint la totalité des caractéristiques militaires espérées et n'a respecté son calendrier Alors que le Royaume-Uni est affaibli par le Brexit- cela a été souligné -et que le partenariat avec l'Allemagne repose aujourd'hui plus sur une affirmation politique que sur une réalité opérationnelle, la situation est extrêmement fragile et inquiétante. C'est un sujet, madame la ministre, qu'il conviendra d'aborder en profondeur avec vous. profondeur avec vous. L'effort particulier du projet de loi dans le domaine du renseignement doit être salué, puisqu'il est susceptible de fédérer des partenaires autour de la France, tout en contribuant à l'autonomie stratégique européenne. De nombreuses questions pourraient être abordées : la réflexion sur le dispositif Sentinelle ; le patrimoine immobilier sur la ville de Paris ; le risque de suractivité qui pèse sur les armées ; et bien d'autres Je laisserai le soin à mon collègue Gérard Poadja, sénateur de Nouvelle-Calédonie, d'aborder les spécificités de cette LPM qui concernent les outre-mer, et notamment la zone Pacifique.

madame la ministre, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des affaires étrangères et de la défense, cher Christian, mes chers collègues, la préparation et le vote d'une loi de programmation militaire sont des moments importants du quinquennat. Il s'agit de définir l'avenir de la défense nationale, donc de la sécurité du pays dans un contexte géopolitique marqué par une instabilité chronique. À l'heure en effet où les grandes puissances s'affranchissent du système onusien en rejetant le multilatéralisme, il est primordial que la France puisse assumer matériellement et humainement la responsabilité inhérente à son rang de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela ne semble possible que si la défense française reste crédible. Pour cela, nous devons fixer et atteindre des objectifs permettant de préserver notre indépendance stratégique. Avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de remercier tout particulièrement le président Cambon pour sa constante implication et sa volonté de travail collectif. Le travail de Le travail de notre commission a permis de compléter le texte du Gouvernement, mais aussi de donner des moyens de contrôle au Parlement, alors même que l'on sent poindre, parfois, une certaine défiance à son encontre. Nous avons ainsi créé les articles 6 et 6 pour être en mesure de vérifier l'état d'avancement et le suivi des livraisons d'équipements. Je me réjouis, madame la ministre, que nos amendements aient permis de progresser sur ces sujets et que nous convergions vers un dispositif. L'amendement que vous nous proposez pour donner le point de passage de la trajectoire d'équipement en 2021 est très important pour le suivi de l'exécution de la LPM. Sur les grands équilibres de la loi, M. Cambon a très bien résumé la situation : l'inflexion et les intentions sont louables, mais les aléas, nombreux. Les risques sont bien présents. Ils pèsent sur l'outil de défense, qui, je le rappelle, ne peut souffrir de ruptures capacitaires, sous peine de subir des décrochages irrattrapables.

Mais des 3 milliards d'euros aussi attendus que nécessaires pour les années suivantes ? Seront-ils au rendez-vous en 2023 ? Les années 2024 et 2025 feront l'objet d'une actualisation prévue en 2021. Or c'est sur ces deux années qu'une partie significative de l'effort devra être concentrée pour porter les ressources des armées à un montant correspondant à 2 % du produit intérieur brut. En définitive, 67 % seulement des besoins sont couverts de manière ferme. Les tableaux de trajectoires financières sont clairs : les deux tiers de l'effort interviendront après l'élection présidentielle de 2022. Le volet que vous appelez « à hauteur d'homme » est profondément fragilisé par l'insuffisance des crédits d'infrastructure. Il manque 1,5 milliard d'euros. En 2025, 60 % des infrastructures de la défense seront considérées comme « dégradées ». Comment préparer l'avenir dans ces conditions ? J'en viens maintenant à la part consacrée aux équipements, qui représente 112,5 milliards d'euros sur la période 2019-2023, soit 22,5 milliards d'euros par an en moyenne, contre 18,3 milliards d'euros en 2018. Cela devrait permettre certaines livraisons anticipées, tel que le programme Scorpion pour l'armée de terre. La Marine nationale devrait bénéficier de nouveaux sous-marins nucléaires- vous l'avez dit -, de FREMM et de FTI d'ici à 2025. L'armée de l'air bénéficiera de nouveaux avions ravitailleurs, de drones et d'avions de chasse nouveaux, vingt-huit Rafale, ou rénovés, par exemple des Mirage 2000 D. Le nombre d'avions ravitailleurs et de transport stratégique est porté de douze à d'ici à 2025 et une livraison des douze premiers exemplaires sera achevée dès 2023. Toutefois, de nombreuses inquiétudes persistent. Le projet de loi que vous nous proposez ne comble pas les lacunes capacitaires. Certaines ne seront même pas résorbées en fin de programmation. des véhicules des VAB seront encore en service ; 80 hélicoptères Gazelle atteindront les quarante ans de service ; seuls 50 % des chars Leclerc auront été rénovés, et leur parc réduit de 17 %. Madame la ministre, pensez-vous que ce soit suffisant pour prétendre jouer un rôle décisif dans la lutte contre le terrorisme ? Est-ce au niveau, à l'heure où la Chine, la Russie et les États-Unis poursuivent une politique d'investissement qui nous donne le vertige ? Mes chers collègues, on ne peut pas aborder les problématiques d'équipements sans revenir un instant sur les procédures d'acquisition de matériels. La réforme de la DGA et l'allégement des requêtes pour les achats en plus petite quantité sont des points positifs. Par ailleurs, et comme dans de nombreux domaines, il apparaît clairement que la France a, une fois encore, surtransposé le droit européen, alors même que la directive 2009/81/CE avait été négociée, pour l'essentiel, sous présidence française de l'Union.

Je souhaite également attirer votre attention sur l'importance de la régénération des matériels. Les opérations extérieures, ou OPEX, et le maintien en condition opérationnelle, ou MCO, sont intrinsèquement liés. Les 22 milliards d'euros consacrés à l'entretien programmé des matériels, soit un montant annuel moyen de 4,4 milliards d'euros, sont bienvenus. C'est 1 milliard d'euros supplémentaires par rapport à la LPM précédente. L'autre défi tient à l'anticipation et à la gestion de l'usure de ces matériels. Cette question est très importante, et il faut travailler main dans la main avec les industriels. Je tiens à saluer l'amendement qui a été adopté par la commission des finances sur proposition de notre collègue Dominique de Legge concernant ce que l'on appelle « les liasses ». Acheter du matériel, c'est bien ; mais s'assurer de la propriété pleine et entière des modes d'emploi, c'est mieux c'est mieux ! C'est vrai ! Cette LPM annonce l'inflexion d'une dynamique très négative. Depuis plus de vingt ans, les dividendes de la paix nous ont incités à baisser la garde ! Cette LPM nous redonne l'espoir de revenir de revenir au niveau qu'exige aujourd'hui la sécurité de la France. Mais nous sommes inquiets quant à la date effective des investissements, qui se concrétiseront pour beaucoup après 2023. L'ennemi de la LPM- chacun le sait -, c'est Bercy. Aucune des dernières LPM n'a été appliquée conformément au vote du Parlement. Le rôle du Sénat doit consister à contrôler sa bonne mise en oeuvre. Je sais, madame la ministre, votre investissement personnel et celui de votre cabinet pour défendre cette LPM. Il nous appartient désormais de vous aider à l'appliquer conformément à nos ambitions à tous, dans l'intérêt de nos armées et de la France. Dès lors, soyez sûre que nous serons au rendez-vous à chaque examen budgétaire, chaque année, mais aussi dès que nous le pourrons, pour vérifier que nos armées disposent des moyens nécessaires à leurs missions. La France ne peut plus se contenter d'effets d'annonce en ce domaine.

que l'a rappelé l'Assemblée nationale, les outre-mer français et les zones économiques exclusives qui leur sont rattachées constituent un enjeu stratégique majeur pour la souveraineté de la France. Il faut veiller au renouvellement des équipements matériels et permettre aux militaires d'exercer au mieux leurs missions dans cette zone. Ce projet de loi a pour ambition de renouveler les capacités opérationnelles et les équipements des armées, notamment par la livraison pour 2025 de six patrouilleurs dans les outre-mer. Je me félicite de cette modernisation annoncée, mais j'ai une inquiétude. Madame la ministre, vous avez indiqué que les deux patrouilleurs assurant actuellement la surveillance de la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie seraient retirés du service actif en 2020. Or les deux nouveaux patrouilleurs devraient être livrés à l'horizon 2021-2022. Comment la surveillance de nos eaux territoriales va-t-elle être assurée durant cet intervalle ? Il serait inconcevable de laisser notre espace maritime en proie aux pillages pendant une ou deux années. Sans patrouilleurs, la souveraineté de la France dans le Pacifique serait mise à mal. à mal. En outre, cette LPM veut améliorer les conditions de travail de nos militaires. Or nous devrions avant tout réduire les inégalités qui persistent entre les militaires métropolitains et ceux qui viennent d'outre-mer et du Pacifique. Les hommes et les femmes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna s'engagent avec la même ferveur, le même courage et le même dévouement que tous les militaires. Pourtant, ils ne peuvent pas prétendre à une prime spécifique d'installation lorsqu'ils sont affectés en métropole. Ils ne bénéficient pas non plus des congés bonifiés, et ils font état d'un réel manque d'accompagnement lorsqu'ils ont besoin de se réorienter professionnellement. Je crois que nos discussions devraient aussi porter sur la réduction de ces inégalités. Le Président de la République a affirmé, lors de sa récente visite en Nouvelle-Calédonie, sa volonté de construire un axe indopacifique fort.

à agir et à nous projeter sur un certain nombre de théâtres de plus en plus difficiles et incertains. Comme je vous l'ai indiqué, je pense que cette loi de programmation militaire sera encore meilleure parce qu'elle aura été travaillée collectivement.

un premier effort tout à fait significatif, de 1,8 milliard d'euros de plus qu'en 2017. C'est tout à fait en ligne avec l'ampleur des progressions qui auront lieu à partir de 2019. En considérant la situation de manière dynamique, on ne peut pas dire que l'ensemble des efforts sont renvoyés à la dernière partie de la loi de programmation militaire. quelques chiffres valent mieux qu'un long discours. Entre 2019 et 2023, la progression annuelle des moyens tels qu'ils sont prévus dans cette loi de programmation militaire est, en moyenne,

donc une marche qui me paraît parfaitement franchissable et réaliste au regard de l'ambition qui est la nôtre. En tout cas, elle est beaucoup moins raide que certains veulent bien l'indiquer.

une fois, ne voyez pas cela comme un risque. C'est au contraire une assurance que nous nous donnons collectivement et que le Parlement, je crois, se donne aussi, à travers ce rendez-vous si important. D'ailleurs, l'article 6 vous permet de bien surveiller cette exécution de la LPM, d'en corriger des variations comme il conviendra.

au développement de moyens autres que la provision pour les OPEX et les missions intérieures. Enfin, c'est l'évidence, cette provision portée à 1,1 milliard d'euros nous permettra permettra d'aborder l'avenir avec moins d'incertitudes, et de réduire la différence entre le montant prévisionnel

Ensuite, il est prévu de renforcer de manière ciblée les effectifs en outre-mer, à raison de 120 postes supplémentaires sur la période de programmation, dont 28 dès l'année 2019. Nous avons également pris la décision de commander et de livrer, dès 2019, un patrouilleur léger pour les Antilles. J'avais eu l'occasion de l'indiquer dans le cadre du débat budgétaire ; je le rappelle, car je crois que cette décision est très attendue outre-mer. Quant à la flotte des patrouilleurs dans son ensemble,

Je suis, pour ma part, tout à fait confiante, sachant l'attachement du Sénat au travail législatif et parlementaire de qualité, à nos armées,

qui a, durant plusieurs années d'exercice au plus haut niveau de l'armée, contribué fortement à la prise de conscience de la réalité vécue par l'armée et de ses immenses besoins financiers.

des dispositions d'actualisation de la programmation militaire pour la période 2019-2025. On peut se féliciter que le texte conforte nos armées, notre modèle de défense, et que les moyens soient en cohérence

Cet allongement donne un triple signal aux acteurs, publics comme privés, de la défense : la prévisibilité, sans laquelle aucun investissement n'est possible, la continuité, pour éviter les rustines comptables, et la crédibilité des décisions publiques, garante de l'efficacité. Le prolongement d'un an permet de faire entrer l'armée dans un cercle vertueux pas d'économies de crédits sans justifications et la volonté d'aller, si nécessaire, vers l'arbitrage pour éviter facilité ou complaisance. En définitive, c'est le meilleur moyen pour imposer la confiance dans les décisions publiques qu'appellent de leurs voeux tous nos partenaires internationaux. militaire nous permettra, à cet égard, de réaliser des investissements lourds, afin de permettre à notre armée de mieux accomplir ses différentes missions. Outre l'amélioration des conditions de vie de nos soldats, qui est une exigence morale, nous serons en mesure de nous confronter aux défis impromptus et aux nouveaux périls qui doivent nous amener à une plus grande liberté stratégique sur le terrain.

3 est un double signal, adressé, en premier lieu, aux adversaires de la France et à nos alliés et, en second lieu, aux armées, qui, après toutes les désillusions des dernières années, s'interrogent et, parfois, doutent. Il fixe les orientations de la politique de défense et les moyens militaires entre 2019-2025 en visant l'objectif des 2 % du PIB en 2025- pensions militaires comprises -, découpés en deux tranches : une hausse de 1,7 milliard d'euros par an entre 2019 et 2022, puis de 3 milliards en 2023. Au total, le budget de l'armée sera de 295 milliards d'euros en 2025, couverts de manière ferme jusqu'en 2023, contre 234 milliards d'euros en 2018. Pour substantielle qu'elle soit, cette ambition n'est ni excessive ni démesurée. Elle correspond à une nécessité. Cet article traduit le passage d'une démarche de réaction à une stratégie d'anticipation. Cet effort vise d'abord, bien entendu, à sécuriser les crédits et les recrutements nécessaires à l'application des engagements du Gouvernement. Pour trouver leur pleine efficacité, ces mesures tendent ensuite à restaurer la disponibilité de nos matériels. C'est la moindre des obligations de l'État de donner en permanence à notre armée les moyens de remplir ses missions à une période déterminée. Nous dresserons alors, en 2021, un premier bilan d'exécution, qui nous permettra également de définir plus précisément

des dérapages, qui ont été relevés par la Cour des comptes. Comme on pouvait s'y attendre, ils ont pour origine les déploiements de nos forces armées sur des théâtres d'opérations extérieures et leur mobilisation en soutien de l'opération Sentinelle, dans le cadre de l'état d'urgence, dispositif qui semble appelé à connaître quelques prolongements, maintenant que les prescriptions de la loi de 1955 sont devenues la règle ordinaire du droit ... Pour l'exécution 2016, selon la Cour des comptes, les crédits de la mission sont passés de 31,83 milliards d'euros hors pensions- les crédits dévolus à cet effet sont, soulignons-le, de 7,83 milliards d'euros -à 33,44 milliards d'euros par le jeu des ouvertures de crédits, des fonds de concours, des reports et transferts de crédits les plus divers.

Dans ce contexte, rappelons tout de même que, pour l'année 2018, nous avons des crédits ouverts pour 34,2 milliards d'euros, c'est-à-dire 760 millions de plus que la dépense officiellement atteinte en 2016. Nous verrons d'ailleurs prochainement si le montant des dépenses fixé pour 2017, soit 32,44 milliards d'euros- 1 milliard de moins que pour l'exercice 2016 -, a finalement été respecté. Ayons en tête les nombreuses opérations dans lesquelles notre pays est engagé - Mali, Syrie, Centrafrique,

Ces ressources ne comprennent pas l'éventuel financement d'un service national universel : celui-ci aura un financement qui ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire. » C'est clair

opère un lissage sur l'ensemble de la période 2019-2025 et évite, en répartissant l'effort plus durablement, la très forte augmentation envisagée pour les années 2023, 2024 et 2025, que l'on appelle communément la « bosse budgétaire Cette nouvelle répartition des crédits permet de concrétiser l'engagement dans la durée, et donc d'éviter les hypothèques qui pèseraient notamment sur le programme 146 relatif aux équipements.

de remettre en cause notre souveraineté financière. En effet, la loi de programmation des finances publiques vise elle-même un autre objectif, qui n'est pas 2 % du PIB pour l'effort de défense, mais la limitation des déficits publics

est défavorable à cet amendement. Je veux enfin rappeler, car c'est la deuxième fois que, avec malice, le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées y fait référence, que, non, nous n'avons pas « raté la première marche ». En effet, malgré l'annulation de 850 millions d'euros, nous avons respecté l'exécution budgétaire 2017.

Cet engagement s'inscrit dans un contexte international qui fait peser une responsabilité particulière sur la France, en tant que membre

avec l'évaluation finale des OPEX. Depuis dix ans, le montant des surcoûts OPEX n'a jamais été inférieur à 850 millions d'euros et dépasse 1 milliard d'euros depuis 2013. Force est de constater que la difficulté à fermer des théâtres d'opérations ainsi que la croissance des risques et menaces dans nos zones d'intérêt conduisent à une augmentation tendancielle du coût des OPEX et, par conséquent, à un décalage croissant avec une dotation initiale. Pour autant, le présent projet de loi ne vise pas à remettre en cause le principe du montant de la provision qui a fait l'objet d'un arbitrage d'ensemble sur la programmation. À cet égard, la provision, portée de 450 millions à 650 millions d'euros dans la loi de finances initiale pour 2018, et qui atteindra 1,1 milliard d'euros en 2020, permet de redonner à la mission « Défense

pose est celle-ci : quand un conflit est-il terminé ? Il suffit de penser à la deuxième guerre américaine en Irak ou à notre intervention actuelle au Sahel ... Il est donc nécessaire d'adapter notre droit à l'évolution des conflits. Je sais qu'une réflexion est en cours ; elle vise à combler une lacune de l'article 35 de la Constitution. Ce dernier oblige le Gouvernement à informer le Parlement, puis à soumettre à un vote la prolongation de cet engagement s'il dépasse quatre mois. Passé ce délai, il ne prévoit aucun bornage dans le temps. Cela avait d'ailleurs été rappelé dans un rapport sénatorial en 2016 par nos collègues Gilbert Roger et Jean-Marie Bockel. La future réforme constitutionnelle nous donnera l'occasion de nous saisir de cette question. François Pillet l'évoque d'ailleurs dans le projet de réforme qu'il a soutenu sur proposition du président Cambon ; il souhaite subordonner la prolongation d'une OPEX à une autorisation régulière en organisant un débat suivi d'un vote. Le groupe socialiste et républicain désire aller plus loin.

ce sera carrément chose impossible. Ma collègue Hélène Conway-Mouret et moi-même avons proposé à la commission de protéger vos crédits contre ces aléas qui désorganisent la politique d'investissement de votre ministère. C'est pourquoi nous avons inséré dans le texte plusieurs éléments en ce sens, dont deux sur lesquels vous entendez revenir à cet article à cet article : la prise en compte du coût de l'usure des matériels dans le calcul du coût des OPEX, le plafonnement de la participation de votre ministère au financement interministériel du surcoût des OPEX. Nous regrettons vivement, madame la ministre, que la position du Gouvernement soit hostile à nos apports. Naturellement, nous ne sommes pas dans le secret des décisions interministérielles, mais nous soupçonnons fortement que le point de vue de Bercy a forgé la position du Gouvernement. Les enjeux de ce texte dépassent pourtant ceux de l'orthodoxie budgétaire et j'émets le souhait que votre ministère puisse peser en ce sens dans les arbitrages budgétaires à venir. C'est toute la question de la crédibilité de la loi de programmation militaire. Si aujourd'hui Bercy commence déjà à nous faire des misères, imaginez ce qu'il va se passer à la fin de chaque année civile !

nous avons beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi le Gouvernement souhaite revenir sur les éléments de sécurisation du budget des armées que notre commission a introduits à cet article. Mon collègue Cédric Perrin, rapporteur comme moi du programme 146, et moi-même avons eu à coeur de mettre les chances de votre côté et du côté de nos armées, face à des logiques de régulation budgétaire à court terme qui peuvent être particulièrement défavorables aux moyens de la défense, lesquels s'inscrivent, eux, dans le long terme. terme. Il est de la responsabilité et du rôle du Sénat de dépasser ces logiques budgétaires court-termistes. Nous nous attendions à ce que vous soyez à nos côtés dans ce combat.

au plus fort de cet interventionnisme, avec pas moins de 33 000 hommes et femmes de troupe, officiers et sous-officiers en état d'alerte et d'intervention. C'est considérable ! À chaque fois, un décret d'avance, gagé sur des annulations et redéploiements de crédits d'autres missions budgétaires, est venu combler l'effet budgétaire de cette externalisation de nos troupes. donc face à une autorisation donnée pour le premier milliard d'euros, avant que nous puissions constater une forme de primauté des dépenses militaires sur toutes les autres, puisque l'affectation des ressources interministérielles resterait acquise au ministère de la défense. En quelque sorte, place Balard, pour la révision des services votés, on repassera ... alors qu'on aurait sûrement eu beaucoup à faire du point de vue des 4,2 milliards d'euros de redevance que nous devrions acquitter à Opale Défense pour disposer de l'Hexagone Balard.

qui fixerait, pour le financement interministériel des opérations extérieures et des missions intérieures, une limite maximale égale à la quote-part du budget du ministère des armées dans le total du budget de l'État.

Tout simplement parce que, comme je l'ai dit précédemment, nous ne sommes plus là dans un débat de programmation : nous franchissons insidieusement la frontière vers un débat sur la gestion des crédits. Or il est d'ores et

est inférieure au montant total des dépenses des OPEX et des missions intérieures, alors un financement interministériel sera mobilisé. À l'inverse, si cette provision s'avère supérieure au montant total de ces opérations, le bénéfice en sera maintenu au ministère des armées. Je veux également dire que, au-delà du débat de principe sur le fait que nous passons de la programmation à la gestion, il ne faudrait pas rigidifier par avance la gestion des crédits de l'État, et ce d'autant moins que, dans la période récente- en 2017, pour ne citer que cette année -, la part du ministère des armées se trouvait être égale dans le cadre du financement interministériel à sa part dans le budget de l'État. C'est la Cour des comptes qui l'indique, puisqu'elle estime que la contribution du budget du ministère à la couverture de 1 milliard d'euros de surcoût au-delà de la provision a été égale à 200 millions d'euros. Or 200 millions d'euros sur 1 milliard, c'est à peu près la part du budget du ministère des armées sur le total du budget de l'État. Je comprends parfaitement votre intention extrêmement bienveillante, mesdames, messieurs les sénateurs, mais je ne voudrais pas que nous anticipions sur une gestion qui n'a pas encore eu lieu et que nous la rigidifiions par principe, car, après tout,

sur les opérations extérieures et intérieures. Tel est le droit actuel. Votre assemblée a souhaité ajouter au périmètre des opérations extérieures et intérieures couvert couvert par la provision non seulement les dépenses du titre 3, mais également les dépenses d'équipement du titre 5.

je veux indiquer que, d'une part, nous avons intégré ces éléments dans notre propre prévision budgétaire et que, d'autre part, si l'on voulait aller dans le sens que le Sénat préconise- c'est-à-dire intégrer les dépenses d'équipement à la provision

la nécessité de ne pas pénaliser le budget des armées par une provision qui serait trop importante par rapport au reste du budget. Pour ces raisons, l'amendement n° 132 vise à à la rédaction initiale du texte, afin de ne pas rendre la provision de 1,1 milliard d'euros, qui est l'objectif que nous souhaitons atteindre en 2020, insuffisante par rapport à ce que nous voulions faire, et recréer ainsi

nous constaterions la suppression pure et simple de la provision pour les OPEX et les missions intérieures. Par conséquent, privés de cette provision, nous serions obligés d'aller puiser dans les autres crédits des armées, ce qui affaiblirait

de la même logique. Le Gouvernement reconnaît en quelque sorte qu'il envisage de faire supporter aux armées l'essentiel du financement interministériel de ces surcoûts.

un amendement d'appel, puisque le sujet, si j'ai bien compris l'argumentaire, est moins la suppression de la provision pour financer les OPEX et les missions intérieures que les pouvoirs respectifs du Parlement et du Gouvernement dans le cadre du déclenchement des interventions extérieures. Il s'agit donc d'un autre débat, institutionnel, qui concerne l'article 35 de la Constitution.

Les surcoûts OPEX excluent en revanche les dépenses liées à l'attrition, c'est-à-dire le remplacement des matériels détruits en opération. » Dois-je en conclure que les matériels détruits en opération n'ont pas vocation à être remplacés et que le financement du remplacement n'est pas assuré ?

annuel. À ce titre, la réforme constitutionnelle à venir devra nous permettre de préciser le cadre d'intervention des troupes françaises et le contrôle du Parlement. Nous l'avons vu avec l'opération menée en Syrie en avril, le cadre constitutionnel en matière d'intervention est suffisamment permissif pour pouvoir se passer du Parlement. Ainsi, si en pratique une déclaration de guerre, une opération extérieure ou une intervention extérieure ponctuelle sont extrêmement proches, les dispositions constitutionnelles y afférentes sont bien différentes. Autre écueil majeur, qui n'est pas l'objet de l'amendement, mais qui doit nourrir le débat, l'intervention extérieure peut commencer sans même une information préalable du Parlement, comme si les récents exemples correspondaient à une prise de décision immédiate du Président de la République, sans préparation. Enfin, j'en viens au fond de l'amendement, le Parlement ne dispose que d'un contrôle tout relatif sur le lancement des OPEX et leur prolongation. Ainsi, le Gouvernement n'est tenu de soumettre au vote du Parlement que la prolongation d'une

Cet amendement s'inscrit dans le droit fil de nos échanges sur la sécurisation des moyens de la loi de programmation militaire.

est celle qui est conforme au programme de stabilité, c'est-à-dire, un cours à 60 dollars, avec une parité euro-dollar de 1,1.

J'ai parfaitement compris l'esprit dans lequel la commission avait travaillé en adoptant un amendement tendant

prend déjà en compte la volatilité des cours du pétrole en prévoyant des mécanismes de couverture contre le risque de fluctuation des cours et en procédant à des achats à terme, à un prix convenu à l'avance, ce qui permet de se prémunir contre une éventuelle hausse des cours. C'est donc un sujet que nous suivons avec beaucoup d'attention en gestion.

à notre rendez-vous de 2021 sur la correcte évaluation des dotations de financement de carburant.

républicain affiche son soutien aux 6 000 postes supplémentaires ; pour autant, nous regrettons une augmentation brutale et hasardeuse ; brutale, car 75 % des recrutements sont prévus après 2023, et hasardeuse, car le réel effort est laissé aux soins des futurs dirigeants. Est-ce cela, la LPM « sincère et réaliste » que souhaitait la Cour des comptes ? La perspective d'évolution des effectifs que nous proposons est plus linéaire et plus adaptée à l'intégration des nouvelles recrues au sein des armées. C'est dès aujourd'hui que nous avons besoin de renforts supplémentaires. Prenons un exemple : la grande majorité des recrutements ira au renseignement et à la cyberdéfense- c'est une bonne nouvelle et nous nous en félicitons -, mais il faut entre deux et trois ans pour former correctement un agent dans ce domaine. Aussi, en décalant la majeure partie des recrutements à la fin du mandat, c'est seulement en 2025

introduire, année par année, la possibilité de contrôler la mise en oeuvre de la future loi de programmation militaire. Si l'on recule encore d'un an son actualisation, on n'ira pas dans le sens souhaité d'un meilleur contrôle du Parlement. L'avis de la commission est donc défavorable.

Conway-Mouret. L'objet de cet amendement est d'inscrire dans le corps de la LPM le dispositif de l'amendement adopté par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, à l'alinéa 196 de l'article 2 du rapport annexé au présent projet de loi. Il s'agit d'assurer l'information du Parlement en amont de ce rendez-vous, sous la forme d'un document préparatoire dressant un premier bilan des efforts consacrés à la remontée du niveau d'activité et définissant des objectifs de progression de la préparation opérationnelle entre 2021 et 2023, puis entre 2023 et la fin de la période de programmation, 2025.

Le Parlement devra disposer en amont de toutes les informations indispensables à cette évaluation et nous considérons qu'il est important que le projet de loi liste et recense clairement les droits à l'information et les pouvoirs de contrôle du Parlement sur son exécution.

le bilan visant la remontée du niveau d'activité des armées est très important pour le contrôle parlementaire. Néanmoins, la commission a une analyse sensiblement différente, dans la mesure où il ne lui paraît pas souhaitable

qu'il ne peut s'agir que des décisions prises avec l'accord de la France. Quel est l'avis de la commission ?

en densifiant les apports stratégiques de la revue stratégique, le support affiché de la présente loi. Ce document, qui évalue les mutations contemporaines de l'espace stratégique, devra prendre en compte les stratégies dites « intégrales » ou « de guerre hors limites

géostratégique pourrait rendre cet exercice utile -, et je n'exclus évidemment pas que cette actualisation de 2021 prenne en compte des éléments de contexte géostratégique que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui.

d'une loi de programmation des finances publiques, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées souhaite retirer le deuxième budget de l'État de l'effort demandé à l'ensemble des services et secteurs publics

Mme la ministre. Cet amendement a pour objet le bilan de l'exécution de la loi de programmation militaire, lequel doit être adossé chaque année au rapport annuel de performance, ou RAP, qui est lui-même annexé au projet de loi de règlement.

Ces informations nouvelles s'ajouteront à celles qui figurent d'ores et déjà dans les réponses aux questionnaires parlementaires transmis annuellement, ainsi que dans les projets annuels de performance et les rapports annuels de performance qui sont annexés aux documents budgétaires,

Cet amendement a pour objet l'élaboration d'un document budgétaire consolidé, qui contiendrait toutes les informations pertinentes dont le Parlement a besoin en vue de la préparation du débat annuel sur le projet de loi de finances. Il ne s'agit pas de proposer une réplique de la VAR, mais d'extraire de ce document ce qui pourrait être utile ce dont les parlementaires auraient besoin pour préparer convenablement le débat budgétaire. À notre sens, la VAR doit faire, à cette fin, l'objet d'un travail commun entre les commissions parlementaires permanentes, les ministères concernés et les administrations.

Dans ce contexte, une mesure performative, telle que l'utilisation des mots « le ou la militaire », peut revêtir de l'importance. Elle peut contribuer positivement à modifier la perception de notre armée. La féminisation de nos armées est récente, et le caractère masculin du milieu militaire explique que les femmes y ressentent davantage que les hommes la nécessité de faire leurs preuves pour s'y imposer, notamment lorsqu'elles y exercent des fonctions d'autorité. En 2015, j'ai été corapporteur du rapport intitulé. C'est l'un des sujets dont nous

visibles les femmes militaires et, ainsi, de défendre et de favoriser la mixité dans les métiers, gage d'amélioration du point de vue tant qualitatif que quantitatif. Quel est l'avis de la commission ?

Or les personnels médico-civils des armées verraient dès à présent leur âge de départ à la retraite reporté de trois

de permettre l'accélération du renouvellement générationnel. En outre, si le corps d'appartenance est le même, les conditions d'emploi, sur certains

Quel est l'avis de la commission ?

que les Français établis hors de France, lesquels ont peut-être plus besoin que les autres d'une formation aux questions de défense, ne soient pas associés à ce processus. Quel est l'avis de la commission ?

et qui constitue aujourd'hui l'article 10 . Cet article vient rehausser l'autorisation d'absence des réservistes à huit jours par année civile, tout en permettant aux entreprises de moins de 250 salariés de maintenir cette autorisation à cinq jours, comme c'est actuellement le cas. Ces dernières années, une véritable dynamique de dialogue et de partenariat s'est dessinée entre le ministère des armées et le monde de l'entreprise. Elle s'est traduite par la signature, à ce jour, de plus de 500 conventions de partenariat, portant à 36 000 le nombre de réservistes du ministère des armées pour un objectif de 40 000 à la fin de 2018. Ces chiffres sont très encourageants pour la montée en puissance de la réserve opérationnelle. Cette logique incitative a l'avantage de conférer aux entreprises la qualité de partenaire de la défense, une visibilité, un logo et un label valorisable. Il paraissait donc difficile de casser cette dynamique. Il aurait même été contre-productif d'instaurer des contraintes trop fortes pour nos entreprises, dont certaines sont très ouvertes à l'égard de la réserve opérationnelle.

Nous soutenons donc le présent article, dans cette rédaction qui nous paraît adéquate et équilibrée, au regard de la réalité du monde de l'entreprise et de cette relation de partenariat que je viens d'exposer. La parole est à Mme Christine Prunaud, sur l'article. L'introduction par nos collègues députés d'un article instituant une autorisation d'absence pour que les réservistes soient libérés de leurs obligations professionnelles en cas de réquisition constitue une avancée importante. Cette disposition permet d'accorder une place de choix à la réserve civile dans le dispositif national civique. Il est toutefois essentiel de rappeler que la réserve intervient en complément des militaires de métier et ne constitue pas une force de remplacement. L'article 10 du projet de loi est donc largement perfectible. Si la mobilisation des réservistes dans une très petite entreprise peut poser de vrais problèmes d'organisation et de fonctionnement à cette dernière, le seuil de 200 salariés initialement fixé me semble peu approprié. Il est paradoxal que, d'un côté, on augmente le nombre de jours d'activité possibles dans la réserve, et que, de l'autre, on ne prévoie qu'une autorisation d'absence très partielle. Comme cela a été dit à plusieurs reprises sur les travées de cet hémicycle, la défense en France est l'affaire de toutes et de tous. Les entreprises doivent donc pleinement participer à cet effort, et les réservistes doivent avoir les moyens de répondre à l'appel qui leur est adressé. Soumettre l'engagement de réserve au bon vouloir de l'employeur revient à imposer aux réservistes de prendre sur leur temps de repos pour participer aux activités de réserve. Cela pose la question de l'efficacité de la réserve, mais également celles de sa vocation et de son caractère de solidarité nationale.

M. Ronan Le Gleut. La rédaction nouvelle proposée pour l'article L. 3142-89 du code du travail prévoit le passage de cinq à huit jours de l'autorisation d'absence octroyée aux salariés des entreprises de plus de 250 salariés au titre de leurs activités de réserve. Or cette hausse du nombre de jours n'a jamais été sollicitée, ni par les réservistes ou les associations qui les fédèrent, ni par le ministère des armées, ni par le secrétaire général de la Garde nationale, bien que ce dernier soit impliqué dans le développement de conventions signées entre l'armée et les entreprises aux fins de favoriser l'activité des salariés engagés dans la réserve. De plus, l'autorisation d'absence au titre de la réserve est dans les faits peu appliquée. En effet, les salariés engagés dans la réserve souhaitent rarement faire état dans leur environnement professionnel de leur engagement dans la réserve pour des raisons multiples et diverses. Le passage à huit jours au lieu de cinq pour pour toutes les entreprises au-delà de 250 salariés s'avère donc inutile et pourrait même être contre-productif, car il pourrait menacer la carrière de certains réservistes ou freiner leur embauche. De plus, De plus, imposer aux entreprises, y compris de taille intermédiaire, des obligations plus contraignantes irait à l'encontre de l'équilibre aujourd'hui acquis et constituerait une contrainte sans doute trop forte pour certaines d'entre elles. Il est donc proposé de supprimer l'article 10 , afin de conserver la rédaction actuelle de l'article L. 3142-89 du code du travail qui semble satisfaire les parties concernées.

À défaut du maintien du système actuellement en vigueur des cinq jours de congé octroyés de droit aux salariés réservistes pour leurs activités au titre de la réserve, il est proposé de réserver ledit congé de droit à huit jours pour les seules entreprises de plus de 5 000 salariés,

classification l'INSEE, comptent de 250 à 4 999 salariés, sont souvent fragiles et leur bon fonctionnement pourrait se trouver affecté, notamment pour les plus petites d'entre elles, par l'octroi obligatoire de huit jours de congé au titre de la réserve.

Quel est l'avis de la commission ?

aucun lien véritable avec la France, qui parfois parlent mal le français et qui peuvent être soumis à des campagnes assez négatives sur la France et ce qu'elle représente. Le présent amendement

la pratique. Dans la pratique, le chef de poste diplomatique a en effet la possibilité de décider d'un report de la JDC dans les pays où l'organisation d'une session peut soit porter préjudice aux personnes convoquées, soit être rendue impossible du fait de contraintes matérielles importantes. En cas de report, c'est le poste qui informe les jeunes de la possibilité de participer à une JDC à leur retour en France si ce retour a lieu avant leurs et leur délivre une attestation provisoire de report permettant de justifier leur régularité au regard du service national français, ne compromettant donc en aucun cas les droits des jeunes concernés.

inconcevable de vouloir supprimer ces JDC qui ne coûtent quasiment rien, sinon peut-être un café et un croissant- et encore, certaines ambassades ne les offrent même pas ! -, alors que l'on va dépenser des millions d'euros pour le service

faciliter les conditions d'exercice des volontaires. Malheureusement, si ces deux types de dommages physiques et psychiques font partie intégrante du dommage corporel, l'évaluation juridique des souffrances psychiques est souvent trop complexe. Concrètement, en cas d'antécédents psychiques, le préjudice risquerait de ne pas être reconnu, la causalité entre l'activité de réserviste et les troubles étant difficilement prouvable. La précision permettrait de permettrait de créer une forme de reconnaissance du fait que l'activité de réserviste peut conduire à des troubles psychiques. Quel est l'avis de la commission ?

M. Ronan Le Gleut. Les Français qui effectuent spontanément une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, ou qui souscrivent un contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle remplissent déjà pleinement leur devoir citoyen. La journée défense et citoyenneté est donc totalement inutile. De plus, exempter ces citoyens libérerait du temps et du personnel d'encadrement pour l'institution. Il s'agit par conséquent d'une mesure de bon sens. Quel est l'avis de la commission ?

Ce secteur d'activité très concurrentiel voit ses besoins augmenter chaque année. Or, contrairement au secteur privé, l'armée reste peu attractive pour les professionnels de l'informatique, cette tendance s'amplifiant d'ailleurs réserve. Cet amendement a pour objet de fournir un état des lieux des professions liées au secteur de l'informatique et, ainsi, de favoriser un recrutement efficient de réservistes voie état-major spécialisés dans le domaine de l'informatique.

et aborde notamment le problème des différents métiers de la réserve. Le recrutement et la fidélisation des réservistes dans le domaine de la cyberdéfense sont évidemment l'une de nos priorités et font l'objet de toute l'attention du ministère, qu'il s'agisse des réservistes opérationnels ou citoyens.

La montée en puissance de la réserve opérationnelle nécessite d'améliorer et de fluidifier le recrutement pour pallier la complexité du processus d'engagement. La réalisation de cet objectif passe par une simplification de la formation initiale des réservistes. L'article L. 4211-4 du code de la défense inscrit la préparation militaire d'initiation ou de perfectionnement comme une voie de recrutement pour la réserve opérationnelle. Toutefois, la préparation militaire est actuellement limitée aux par l'article L. 115-1 du code du service national Cette limite d'âge complexifie beaucoup le recrutement des réservistes de plus de trente ans et prive ainsi le ministère des armées d'une partie du vivier des réservistes âgés de trente à quarante ans.

Quel est l'avis de la commission ?

Fort heureusement, de plus en plus d'étudiants s'engagent ou souhaitent s'engager et servir dans la réserve. Mais si l'engagement associatif est souvent valorisé par l'université, ce n'est pas le cas de l'engagement dans la réserve opérationnelle. L'étudiant réserviste peut même être sanctionné en cas d'absence, dès lors que cette absence ne constitue pas un motif légal d'aménagement ou de rattrapage du temps universitaire. La décision reste donc toujours à la discrétion du professeur. Les étudiants réservistes ont besoin d'un parcours aménagé qui reconnaisse le réserviste étudiant et la réserve étudiante. Il faut légiférer pour que ce parcours soit reconnu dans l'enseignement supérieur. Tel est l'objet du présent amendement.

: La parole est à M. Joël Guerriau. Avec la suppression du service militaire, le monde de la fonction publique se trouve coupé du monde militaire. Pour la haute fonction publique, issue de l'ENA notamment, cela conduit à un éloignement de la réalité quotidienne de la condition militaire et de la défense nationale, alors que certaines décisions structurantes en la matière impliquent l'administration. Pour le monde militaire, cela signifie se priver d'un vivier de talents dont les compétences administratives, techniques ou d'encadrement pourraient être utilisées à profit : l'engagement de jeunes élèves fonctionnaires stagiaires dans l'encadrement du futur service national universel pourrait, par exemple, être envisagé. Plus largement, cet amendement vise à engager une réflexion sur la formation des élèves fonctionnaires en lien avec le monde militaire, et ce dans un souci de rayonnement des armées, de sensibilisation des hauts fonctionnaires à la défense nationale et d'utilisation par les armées de compétences extérieures, lors d'une période de stage, par exemple. Une articulation de ce dispositif avec la réserve opérationnelle pourrait également être étudiée. Quel est l'avis de la commission ?

et à simplifier les démarches individuelles entreprises par les étudiants qui sont engagés dans la réserve opérationnelle. Par ailleurs, dans le contexte actuel de réflexion sur

l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et d'assimiler les périodes de congé de longue maladie et de congé de longue durée pour maladie à des services militaires effectifs, afin de les prendre en compte dans le calcul de la décote « carrières courtes ». En effet, aujourd'hui, ces congés de longue maladie et de longue durée pour maladie sont attribués après épuisement des droits de congé maladie pour des affections graves et invalidantes. La durée de ces congés n'est actuellement pas prise en compte pour la mise en oeuvre du mécanisme de minoration des pensions des militaires qui ont effectué une carrière courte. Cette situation est difficilement

Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement vise à offrir à un militaire réformé à la suite d'une blessure reçue dans l'accomplissement de sa mission opérationnelle la possibilité d'être reclassé dans un emploi civil de son armée d'appartenance. Le nombre de blessés dans les forces armées et dans la gendarmerie nationale a considérablement augmenté depuis trente ans. En parallèle, les gouvernements successifs ont procédé à des substitutions de militaires par des civils pour des postes de soutien et d'administration dans les armées et la gendarmerie nationale. le commandement dispose donc de moins en moins d'emplois d'environnement lui permettant de reclasser ses subordonnés souffrant d'inaptitude. Faute de solution satisfaisante, certains reclassements s'opèrent dans les unités opérationnelles, obérant la capacité opérationnelle de l'unité et aggravant la charge de travail des autres militaires. Pour d'autres encore, la réforme conduit au chômage, compte tenu des difficultés de reclassement.

Quel est l'avis de la commission ?

un reclassement limité à la seule armée d'appartenance du militaire réformé. Par ailleurs, compte tenu de la nature de certaines blessures ou affections qui peuvent en découler,

Le rapporteur l'a rappelé, le militaire dont l'inaptitude entraîne une réforme pour raisons de santé peut d'ores et déjà bénéficier de nombreux dispositifs d'accompagnement, dont le congé de reconversion, l'accès aux emplois réservés ou l'accès à la fonction publique. Bref, il existe de très nombreux dispositifs qui ont vocation à permettre cette reconversion, mais sur un périmètre beaucoup plus large que celui de l'armée d'appartenance. Ces mesures de reclassement sont souhaitables et souvent souhaitées

des missions qui leur sont confiées. Ils subissent de nombreuses blessures et des chocs émotionnels importants qui nécessitent un suivi médical. Compte tenu du nombre croissant de ces missions, ici ou ailleurs, les équipes soignantes sont en nombre insuffisant. Quel est l'avis de la commission ?

Il m'a été répondu en commission que mon amendement était satisfait par les règles applicables au traitement des dossiers individuels, en vertu de l'article 8 de la loi Informatique et libertés, qui dispose : « Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. » Est-ce pourtant aussi simple ? L'article 13 de la loi du 13 juillet 1983

Certains militaires de carrière peuvent quitter l'institution en bénéficiant d'une pension afférente au grade supérieur, ce qui leur permet de disposer d'un indice de rémunération de grade supérieur à celui qu'ils détiennent lors de leur radiation des cadres. En l'état actuel de la législation, ils ne peuvent servir dans la réserve opérationnelle, sous peine de perdre le bénéfice de leur retraite. Cet amendement vise à permettre à ces militaires expérimentés de continuer à servir dans la réserve tout en conservant les avantages de leur pension afférente au grade supérieur. Quel est l'avis de la commission ?

Les zones de défense ont été créées par le décret n° 50-1189 du 29 septembre 1950 relatif à l'organisation de la défense en surface du territoire métropolitain, pour regrouper alors plusieurs régions militaires. Le nombre de ces zones a été fixé à quatre par le décret n° 51-742 du 13 juin leur rôle a été redéfini par le titre IV de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

du service militaire adapté qui existe en outre-mer depuis 1961. Cet amendement est une nouvelle tentative pour permettre aux Français de l'étranger de bénéficier de ce service militaire volontaire, qui, ayant connu un réel succès pendant sa période d'expérimentation, a été prolongé et adapté par la loi du 28 février 2017.

ailleurs, le SMV n'a pas la même vocation que le futur SNU, comme nous le rappellerons lors de l'examen de l'article 2, précédemment réservé. Il est difficilement compréhensible que certaines avancées souhaitées par les sénatrices et les sénateurs soient renvoyées à de futurs projets de loi dont l'examen n'est pas encore programmé. Rien n'empêchera d'intégrer des dispositions de coordination dans des textes à venir. Vous conviendrez qu'il faut s'efforcer d'harmoniser l'accès aux différents dispositifs à vocation citoyenne pour tous les Français. C'est un signal important à donner

pour explication de vote.